La séance est reprise. L'ordre du jour appelle une déclaration du gouvernement suivie d'un débat en application de l'article 50 tirée. De la Constitution relatives à la politique. Bonjour, la France en Afrique. je vais immédiatement donner la parole à Madame, Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Ministre. Vous avez la parole. Monsieur le président. Monsieur le président de la commission des affaires étrangères de la Défense et des forces armées. Mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. Nous le savons tous, les uns et les autres. L'Afrique est une région où se joue une partie de notre avenir commun. Ce constat qui avait fait le président de la République en 2017. Devant les étudiants de l'université de Ouagadougou reste résolument actuelle. Nous partons d'une réalité, l'Afrique subsaharienne compte aujourd'hui un milliard 100 millions d'habitants et selon les Nations-Unies. Sa population devrait doubler d'ici 2050. L'Afrique c'est donc un dynamisme réel dans notre voisinage immédiat avec ce que cela signifie en termes de défis comme en termes d'opportunité. Du côté des opportunités. Ce sont des perspectives de développement avec une participation toujours plus importante du continent dans dans l'économie mondiale. Ce sont des marchés à consolider ou investir pour nos entreprises. C'est une jeunesse. Dynamique entreprenante créative. Côté défi ce sont tous les risques induits précisément par cette forte croissance démographique dans un espace très exposé par ailleurs au changement climatique et à ses multiples et terribles conséquences. Tout cela nous met face à des enjeux immenses concernant le développement la transition climatique. Le partage de la richesse, l'éducation ou encore la santé avec toutes les conséquences possibles sur les plans sécuritaire sanitaire migratoire et pour toutes ces raisons et devant toutes ces réalités, nous avons bel et bien selon une formule employée par le président de la République. Fin février un destin lié avec le continent africain. Ce n'est, je le toujours ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, c'est un fait et tout dépendra de ce que nous en faisons. On a trop souvent considéré de ce côté de la Méditerranée que les relations entre la France et l'Afrique était. Un peu comme celle de Montaigne et La Boétie parce que c'était lui et parce que c'était moi. Nous avons trop longtemps pensé que nos relations aller de choix en faisant comme si les Africains ne donnerai toujours leur préférence et depuis longtemps. C'est un réflexe. Immuable qui nous est venue, or rien n'est plus faux. Et dans un monde toujours plus concurrentiel. Cette attitude conduirait inévitablement à perdre en crédibilité au moment précis où notre coopération commune n'a jamais été aussi souhaitable. L'époque où certains considérer l'Afrique comme le terrain d'une rivalité à somme nulle entre puissances est également totalement dépassé. Les pays africains ont depuis bien longtemps diversifier leurs partenariats, comme nous tous d'ailleurs. En somme, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, la politique étrangère de la France en Afrique c'est mettre fin définitivement à cette logique et cette mentalité de l'évidence pour mieux avancer ensemble, main dans la main en véritable partenaire. nous avons pour cela des atouts nombreux et des atouts qu'il nous faut faire valoir. Le 1er de ses atouts, c'est l'intensité de nos Liens humains. C'est cette langue française que nous partageons avec l'Afrique francophone ces ce millions de Français de la Réunion et de Mayotte qui vivent en Afrique et dont nous voulons renforcer l'intégration régionale. Ce sont aussi nos diasporas aussi bien les Français qui vivent en Afrique que les Africains qui vivent en France. Sans oublier bien sûr ces millions de nos compatriotes qui sont liés à ce continent. Et enfin il y a l'ambition de la France, la France, qui entend donner la pleine mesure de ses moyens à son action. Une ambition qui se retrouve d'abord dans d'aides publique au développement et je voudrais rappeler qu'elle est passée entre 2017 et 2022. De 10 à 15 milliards d'euros par an. La France est ainsi devenu l'an dernier le 4ème bailleur mondial est le seul à avoir accru ses financements sur le continent africain avec plus de 5 milliards d'euros, 5,2 milliards. De financements bilatéraux et multilatéraux destinés à l'Afrique. Et à Bruxelles également au plan européen, nous défendons la place de l'Afrique comme première région de notre solidarité européenne. À une échelle plus globale. Le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Les 22 et 23 de ce mois vise également à conjurer un risque de fracture croissante entre le Nord et le Sud. En voulant répondre aux besoins des pays en développement pour financer notamment la transition écologique et la sortie de la pauvreté. Notre ambition c'est aussi celle-là que nous manifestons en soutenant les attentes de l'Afrique d'être mieux intégrés à la gouvernance mondiale. Nous sommes vous le savez depuis longtemps réseau du Mans, favorable à une réforme du Conseil de sécurité des Nations. de sièges d'un siège pardon de membre. Permanent à un pays africain ainsi. Que nous sommes favorables à une participation pleine et entière de l'Union africaine au G20. Notre ambition, nous la déployons aussi dans notre réseau culturel grâce à 28 institut français et 109 Alliances françaises. Rien qu'en Afrique subsaharienne. Les 108 établissements scolaires affiliés à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger présent sur le continent africain. Sont un autre outil de rayonnement auprès des générations futures. En France, nos universités accueillent un nombre toujours croissant d'étudiants africains. Ils étaient 150.000 en. 2021. En augmentation de 40% par rapport à 2017. Notre ambition, elle se déploie aussi évidemment sur le terrain économique. Et il faut d'ailleurs se méfier de certains faux-semblant, je voudrais revenir brièvement. Les économies africaines s'étant largement mondialisée. Oui, nos parts de marché ont pu marquer le pas. Mais la croissance africaine a été telle que notre présence économique a augmenté en volume avec de plus en plus de PME françaises qui se tournent vers le continent. En 15 ans le nombre de filiales d'entreprises françaises en Afrique a doublé. De même que nos investissements. La France est aujourd'hui le 2ème investisseur étranger en Afrique. Voilà des choses que l'on dit, où l'on lit trop peu souvent. Notre réseau diplomatique est pleinement mobilisée pour soutenir cette dynamique en assumant pleinement nos intérêts. Cette ambition, elle se déploie aussi dans un dialogue continu approfondies avec nos partenaires africains sur tous les sujets d'intérêt commun et ils sont nombreux je voudrais en citer quelques-uns. Au 1er rang de ceux-ci figurent bien sur la lutte contre le changement climatique. En 2021, à la COP 26 de Glasgow. Nous avons ainsi pu être précurseur en nous engageant dans le partenariat pour une transition énergétique énergétique juste les femmes jettent pis pour l'Afrique du Sud pour faire progressivement sortir ce pays de sa dépendance au charbon. Afrique du Sud où je me rendrai d'ailleurs dans deux semaines. Dès le début de la guerre russe en Ukraine. Qui a nous le savons tous très sévèrement aggraver l'insécurité alimentaire est touché en particulier le continent. Nous nous sommes mobilisés en faveur des pays les plus vulnérables. En particulier en Afrique. Nous avons notamment financé et faciliter l'envoi de céréales et l'amélioration de la sécurité alimentaire, comme récemment avec les 20 millions de tonnes d'engrais. Vers le Malawi. Mais j'ai pu me rendre aussi en Éthiopie, où nous avions. Acheminé avec l'aide de l'Allemagne. 26.000 tonnes, si ma mémoire est bonne de céréales à destination du programme alimentaire mondial. Nous avons doublé notre contribution celui-ci et nous travaillons aussi au renforcement des systèmes alimentaires en Afrique. D'un autre côté, la Russie quant à elle et exerce un chantage. Constant sur la reconduction de l'initiative pour l'exportation des céréales par la mer Noire l'accès. Une initiative. Vous vous entendez bien la guerre. En Ukraine est au coeur de nos discussions avec nos partenaires africains. Pour en limiter les conséquences néfastes pour eux j'en évoquer quelques aspects mais aussi. En soi, par ce que l'agression d'un pays souverain par un pays voisin. Est une agression aussi contre les principes fondamentaux de la charte des Nations unies comme le principe de l'égalité souveraine et comme le respect de l'intégrité territoriale des États. Et sans le respect de ces principes. Les États ne peuvent avoir. Ni paix ni stabilité, nous le faisons valoir à l'ensemble de nos partenaires dans le monde entier. Et notamment. Auprès de nos partenaires africains qui parfois ne le voit pas suffisamment voyant l'Europe comme trop loin. Dans notre dialogue avec eux, nous défendons donc sans relâche. La nécessité de maintenir et même d'accroître la pression sur la Russie pour faire en sorte que son agression échouent. Car en réalité, c'est bien. L'avenir L'avenir et la sécurité de toutes les nations souveraines qui est en jeu. Une agression qui serait récompensé. Ouvrirait la voie à d'autres agressions. Là ou ailleurs et donc, tous doivent en être conscients, parce que tous nous sommes concernés. Ce rappel est d'autant plus. Indispensable au moment où 6 chefs d'état du continent, vous le savez s'apprête à se rendre à Kiev et à Moscou dans le cadre d'une initiative de paix dont les contours restent à dessiner. Toute initiative doit s'appuyer sur le plein respect des principes fondamentaux de la charte. Plus généralement, et partout sur le continent, la France, mais sa diplomatie au service de la paix, en Afrique de l'Ouest où les pays du Sahel et du Golfe de Guinée font toujours face à une importante menace terroriste mais je laisserai le soin Ministre des Armées de revenir avec vous mesdames et messieurs les sénateurs, plus en détail sur les aspects militaires de notre action, bien évidemment. Au Soudan, nous sommes en contact avec les 2 parties au conflit. Ce qui nous a permis non seulement d'évacuer des Français désireux de quitter Khartoum. Au mois d'avril ainsi que de très nombreux ressortissants étrangers. Mais. Qui. Sont des contacts qui doivent nous conduire à les convaincre. De renouveler la trêve de la rendre effective est également de rechercher une solution politique qui est nécessaire. Dans les Grands Lacs. Également notre diplomatie tu aussi à la manoeuvre pour soutenir le processus de paix. Enfin nous dialoguons en permanence. Sur les sujets. Est entré à l'état de droit, la démocratie, la lutte contre la peine de mort. L'égalité entre les femmes et les hommes, les droits des personnes LGBT, plus la liberté d'expression ou plus généralement sur l'ensemble des sujets sur lesquels la France a des positions à tenir et d'ailleurs c'est ce que nous faisons. Partout dans le monde que notre interlocuteur soit africain ou non. Car l'autre grande clés de compréhension de notre politique. Qu'étrangères en Afrique. Et as trouvé dans cette volonté clairement exprimée. De bâtir une relation nouvelle équilibrée réciproque et responsable et je cite là aussi les mots du président de la République. C'est exactement ce type de relation que nous menons avec chacun des 54 pays du continent dans le cadre de 54 relations bilatérales. Il n'y a pas une Afrique il y a beaucoup d'Afrique et nous avons 54 partenaires en Afrique. Tous ces pays ont leur spécificité, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne faut pas réduire les relations franco-africaines. Une seule situation au prix de raccourcis, de simplifications comme on en voit tant étant. Se laisser prendre au piège de fausses panique déclinistes ou s'enfermer dans des complexes qui n'ont pas lieu d'être, c'est ne pas être à la hauteur de, de ce qui se passe réellement sur le continent au concrètement. La très grande majorité des cas, nous avons des relations qui fonctionne bien et qui portent leurs fruits. Pour autant, on le sait, il y a aussi des vents contraires et. Nous sommes déterminés. À y faire face. Je pense en particulier à la diffusion de discours anti-français dans certains pays, en particulier dans certains pays d'Afrique francophone. Alors ces discours, nous devons en comprendre l'origine. Ils sont pour partie liée à l'héritage de l'histoire pour partie aux frustrations de la jeunesse et pour partie, nous le savons tous. Également à des entreprises hostile. Souterraine au moins souterraine venant notamment de la Russie et face à chacune de ses raisons à chacune de ces causes. Nous agissons résolument. C'est notamment le sens de notre présence sécuritaire en Afrique avec une dynamique qui est désormais plus partenariale moins visible et là aussi je laisserai le ministre-désormais détaillé notre nouvelle posture. C'est aussi le sens de la démarche entreprise auprès de certains pays où notre relation doit faire face à une mémoire troubler un passé qui ne passe pas. Parce qu'on n'a pas. Assez tôt. Ah résolument en fourni les efforts qui était attendues de nos partenaires africains et qui était, nous le pensons Alors ça a été fait au Rwanda notamment. Un exemple qui doit nous montrer la voie au Rwanda, où nous avons pu mener. Des travaux avec les historiens des 2 pays ce qui a permis à la France de regarder. Notre histoire en face et de mieux construire une relation de confiance. C'est également, vous le savez la voie que nous prenons au Cameroun depuis l'été dernier avec l'installation toute récente d'une commission d'historiens et d'artistes français. Et camerounais et plus globalement, nous donnons un nouveau tournant notre communication en l'orientant davantage vers la jeunesse à laquelle nous voulons montrer la réalité concrète de notre coopération. Derrière ces discours bien souvent inexacts. Je suis redonnée mesdames messieurs les les sénateurs à nos ambassades en Afrique, les moyens de mener elles-mêmes directement les petits projets avec. Des décisions plus rapides, plus visible, plus proche du terrain et des bénéficiaires. Il en va là aussi de notre influence et je vient ainsi de lancer à fond, équipe, France, doté de 40 millions d'euros. Pour certains, cela peut paraître peu mais pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est beaucoup et pour nos ambassades s'est apprécié font équipe France ce qui permet à nos ambassades de monter des projets à haute valeur politique et sur décision rapide, je le redis. J'ai également lancé en début d'année un fond d'appui à l'entreprenariat culturelle avec 20 millions d'euros avec nos ambassades en Afrique puisse directement soutenir les acteurs des industries culturelles et créatives avec lesquelles nous avons tant à faire, et souvent qui ont tente à nous apprendre assez de fonds. Sont complémentaires évidemment de l'action structurante et de plus long terme que mène notre Agence française de développement. Sur le plan culturel. Après la saison Africa. 20 20. Nous inaugureront bientôt à Paris une maison des mondes africains afin de faire rayonner les cultures et les créations africaines en France, mettre en valeur nos diasporas et faire la démonstration que la France et ses partenaires africains sont plus fort et plus influent lorsqu'ils s'unissent. Cette intimité culturelle entre la France et l'Afrique doit aussi nous permettent de rayonner au-delà de nos pays et vers le monde entier. Partout dans le monde, nos instituts programme désormais des artistes africains ou des créations franco-africaines et souvent avec un très grand succès. Et plus que jamais. Nous travaillons avec les acteurs de la société civile avec les entrepreneurs, les artistes, les intellectuels du continent la fondation de l'innovation pour la démocratie. Lancée en octobre dernier avec Achille Bembé. Que je verrai bientôt en Afrique du Sud, puisque je m'y rends. Entend ainsi. Mettre en réseau toutes celles et tous ceux qui inventent, chaque jour des nouvelles formes de vie démocratique sur le continent et tout cela sans donner de leçon avec. Humilité mais aussi avec conviction, nous devons les aider. Nous devons nous appuyer sur. Enfin. Face au défi des manipulations de l'information de la part de puissances déstabilisatrices on est. Au moins une. Nous nous dotons de moyens d'agir. vais augmenter les moyens du ministère en matière de communication et de rayonnement. Et ce mouvement a vocation à se poursuivre. Nous avons ainsi mis en place des dispositifs de veille de détection des manoeuvres hostiles et de riposte en particulier sur les réseaux sociaux. Nous soutenons en parallèle les fact-checkers pardon du franglais que j'utilise et les écosystèmes médiatique africain pour qu'il y ait une presse de qualité et professionnel et j'ai demandé à nos ambassadeurs d'adopter une communication plus offensif, plus visible. nous avons également mener un travail de refonte de la communication de tous nos opérateurs afin que sur le terrain. Bientôt il n'y ait qu'un seul drapeau et qu'une seule équipe France. Voilà, Mesdames, et messieurs les sénatrices et sénateurs avant de passer la parole au ministre des armées. Je voudrais clore mon propos en insistant une dernière fois sur l'un des principaux atouts du continent qui est sa jeunesse. Une jeunesse exigeante. Entreprenante. Fière. Jeunesse qui est résolument ouverte sur le monde. Qui ne veut pas qu'on lui dit ce qui est bon pour elle ou ce qui n'est pas bon, qui ne cherche pas à ce qu'on agisse à sa place, mais simplement à ce qu'on s'investissent dans ces projets dans un esprit de partenariat dans un esprit gagnant gagnant. Une jeunesse en fait qui ressemble tellement à la nôtre. Et une jeunesse qui nous lance un défi, celui de nous renouveler. De changer notre manière de faire et nous entendons cette demande. Le programme de transformation. Nous avons lancé. Je peux vous assurer que tous nos diplomates en Afrique le font vivre avec conviction avec enthousiasme. Et c'est ainsi. Je le sais que la France restera un partenaire. Proche. Pertinent. Fiable de ce continent, continent qui est appelé à occuper une place tellement centrale dans les équilibres du monde de demain. Je vous remercie. La parole est maintenant. Au Ministre. Monsieur Sébastien Lecornu. Monsieur le Ministre de la parole. Merci monsieur le président du Sénat, monsieur le président de la commission des Affaires étrangères. Et des forces armées du Sénat, Mesdames, messieurs les sénateurs. Qu'il me soit permis de revenir plus précisément sur effectivement la la situation sécuritaire et de par là même la question de la présence militaire. Française dans le continent africain. Comme l'a dit la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. L'Afrique était un continent, il y a autant de diversité de situation et sécuritaire et. D'organisation de nos forces armées qui n'a de partenaires. Si je devais dire au fond 5 choses et peut-être après laisser davantage de place au débat à la discussion et permettre enfin de de séances de répondre à l'ensemble de vos de vos interrogations commentaire ou réflexion vous ne manquerez pas de de formuler je pense 5 choses à dire importante sur ce débat. Première déjà si on devait être. Un peu schématique ou caricaturale, au fond, on est en 2023, il y a eu de grandes périodes depuis le début des années 2002 1002, Beaucoup d'intervention française au fond sur fond de de culture d'interposition ou de missions de maintien de la paix dans le cadre des Nations-Unies. Je pense que la plus connue, c'était évidemment l'opération. Licorne c'est toute l'action de la France a mené évidemment. En ainsi en république de Côte d'Ivoire pour faire vite, il y en a d'autres. 2012 1020. Une autre étape, une autre période marquée par la lutte contre les groupes armés terroristes avec évidemment les opérations. Au Sahel notamment Serval. Puis Barkhane décidée par le président de la République François Hollande à la demande des partenaires et notamment du partenaire malien pour lutter contre un certain nombre de groupes armés terroristes avec évidemment des ramifications qui pouvait se faire sur la sécurité sur le sol européen mais aussi sur des menaces plus en 2 jeunes sur lequel je reviendrai dans un instant. J'aimerais le dire sur ces dernières mission Serval comme Barkhane. Ce sont des succès militaires et j'entends ici ou là, parfois des commentaires ou des propos se lever autant qu'il y a pu y avoir des limites politiques à ses interventions en tant que telle sur le terrain tactique sur le terrain militaire, ce qui a été demandé aux forces armées françaises a été marquée par le sceau du succès ou alors que celles et ceux qui portent la contradiction sur ce sujet soit en capacité de nous le démontrer et je le dis puisque ce narratif la il me semble contraire. Aussi au sacrifice des 53 soldats qui sont tombés au Sahel 9 pour faire valent hein trop souvent oubliés pour épervier et 43 pour Barkhane et Monsieur président du Sénat, Mesdames, messieurs les sénateurs qu'il me soit permis d'avoir une pensée particulière pour pour eux, pour leur famille et aussi pour l'ensemble des blessés dans le cadre de ces opérations puisque l'armée française est une armée d'employes qui prend sa part de risques, c'est le moins que l'on puisse dire est que pour le coup, la mission a été a été de ce point de vue un succès, même si elle fut douloureuse. La réalité c'est que. Par le temps, nous avons fini par nous substituer aux différents pays qui parfois nous avait demandé ces interventions et je comprendrais ce point dans un instant pour tirer un certain nombre de conclusions sur ce que nous sommes en train de faire, ça c'est la première des choses. La 2ème des choses c'est de voir aussi que les menaces évoluent elle change et que Paris doit le voir je suis frappé là aussi de voir dans beaucoup de. Commentaires qui peuvent être. Produits ici ou là, y compris dans la presse et de voir au fond que déjà la menace terroriste. Elle a elle a fondamentalement évolué. parfois plus fragmenté, elle en est donc pas moins dangereuse parce que comme elle est plus fragmenté. Elle se balkaniser. Énormément. Elles se, elles sont aussi devient beaucoup plus diffus sur l'ensemble de la, de la zone. Elle est donc aussi plus endogène plus tribal et plus compliqué parfois à renseigner à détecter et à saisir saisir 2ème des choses évidemment qui change, et la ministre l'a dit. Dans le constat qu'elle a qu'elle a très justement formulé c'est que au fond le continent africain. Il s'est ouvert. Il s'est ouvert pour le meilleur comme pour le pire, si j'ose dire. Il s'est ouvert déjà. Un certain nombre. De de diversification et donc au fond des influences qui sont légitimes. Ce sont des États souverains qui ont donc eux aussi choisi de diversifier leurs partenariats de faire jouer au fond une forme de mise en concurrence, notamment sur les questions économiques parfois sur les sujets sécuritaires et compris d'ailleurs capacitaire en matière d'équipement militaire et donc ça évidemment ça nous porte un défi c'est au fond d'être plus attractif vis-à-vis de partenaires qui sont des partenaires ancien pour lequel il y a souvent une relation qu'on pourrait qualifier d'affective et pour cause. Mais pour autant nous avons parfois été très déceptif dans la manière justement d'interagir avec d'autres compétiteurs et puis enfin, évidemment il y a d'autres influences qu'on pourrait qualifier elle de moins. Bienvenue au fond parce que sur fond de compétition économique et évidemment aussi sur fond d'initiatives sécuritaires ou informationnelle. On ne peut pas ne pas citer le compétiteur stratégiques russes en la matière, c'est évidemment la question de Wagner. Mais au-delà de ça, d'autres sujets pourraient être pointée et puis le 3ème élément qui ne fait jamais l'objet de de d'une réflexion me semble-t-il. À Paris, dans les, dans les cercles politiques et intellectuels think tank diplomatique ou institutionnelle, c'est évidemment de voir que le continent africain lui-même est soumis au fond à la tension entre les modèles dit autoritaire d'un côté et de démocratie libérale, de l'autre. C'est quand même la réalité de ce qui s'est passé au Mali et c'est toute la question évidemment des juntes militaires ou au fond dont on constate qu'elles arrivent on reprocherait presque à Paris, le fait qu'elles arrivent et en même temps si on avait dû y faire quelque chose, on nous aurait reproché une forme d'ingérence ou une manière de faire de la politique en Afrique comme jadis c'est-à-dire en intervenant dans les processus soient démocratique soit non démocratique, moi je pose la question devant la Haute Assemblée. C'est un point de réflexion important y compris pour les forces armées compris pour d'autres services qui relèvent de ma tutelle c'est évidemment de se dire, au fond, non seulement il faut renseigner, il faut détecter j'en dis pas plus ici. Dans le cas de la DPR de délégation parlementaire pour le renseignement. J'ai répondu à un certain nombre de questions sur ces sujets et sur ces modifications profondes dans ces pays, ces derniers temps mais enfin au-delà du renseignement au-delà du militaire. Il y a aussi un combat plus politique que sont aussi les valeurs de la démocratie au fond si on devait cité à cette tribune Tocqueville et les grandes valeurs de liberté, au fond, est-ce que c'est un modèle qui convient ou est-ce que c'est un modèle qui ne convient pas cette question auxquelles d'autres continents sont évidemment confrontés l'Afrique évidemment ne y fait pas. Autre aspect important où on est l'état de notre présence militaire puisque là aussi on a un certain nombre de de constats qui sont format formulées dans la presse mais qui sont pas toujours d'une grande exactitude au fond la trois familles de bases militaires différentes en fonction des missions. La première famille c'est au fond le duo Sénégal Gabon. Base avec des éléments prépositionnés depuis désormais très longtemps au fond depuis l'indépendance depuis la conclusion des premiers traités de défense qui sont des pôles de coopération qui à la fois qu'on prenne des accès à des infrastructures qui sont d'ailleurs souvent civils rarement militaire mais qui peuvent être utilisées pour nous à des fins militaires, beaucoup d'offres de formation évidemment pour le partenaire. En tant que tels le Gabon ou le Sénégal, mais aussi pour les mais aussi pardon pour les pays qui sont alentour, c'est encore plus vrai d'ailleurs pour les éléments français positionnés au Gabon dans lequel on a pratiquement 8 à 9 pays autour du Gabon qui peuvent profiter des offres de formation telles que nous les. Organisons là-bas ce sont plutôt des longs séjours. Je rappelle que ce sont des bases dans lequel il n'y a pratiquement aucun armement si ce n'est quelques armements pour pour organiser de la formation si au Sénégal, au Gabon, il doit y avoir un ou 2 VAB par. C'est bien évidemment le le le le le maximum que l'on puisse y trouver la 2ème famille ce sont des bases opérationnelles. Pour le coup de de qui sont dans les classes les plus importantes, c'est évidemment les forces prépositionnées en Côte d'Ivoire à Abidjan Port-Bouët et évidemment la base de Djibouti. Port-Bouët globalement classe 1000 hommes ne 150 personnes pour être précis, Djibouti, on est sur une classe à 1700 personnes. Djibouti à la fois c'est une base pour évidemment. L'Afrique de l'Est on l'a bien vu récemment avec l'opération sagittaire avec l'évacuation des ressortissants à Khartoum s'est Djibouti évidemment qui a été appelé C'est aussi une base évidemment de sécurité pour le partenaire djiboutiens avec des accords de défense et des clauses de sécurité qui sont inscrites. Mais enfin c'est aussi bien sur une base qui est très largement ouverte sur l'indo-Pacifique avec évidemment son accès Naval. Les enjeux de sécurité sur Ormuz Babel Mandel et sur l'ensemble de l'océan Indien connecté en cela cela avec nos éléments prépositionnés aux Émirats arabes unis et bien évidemment dans les phases de Mayotte et de la réunion donc Djibouti à la fois un rôle tourné vers l'Afrique mais en même temps aussi tournée vers l'ensemble de la zone indopacifique c'est de base opérationnelle. Au-delà du fait qu'elles sont importantes par leur empreinte. Elles sont surtout marquées par le fait qu'elles sont de véritables points d'appui au combat et qu'à la différence pour le coup des forces qui sont au Gabon et au Sénégal, là on a des forces qui combattent qui peuvent être engagés à la demande du président de la République, en fonction aussi évidemment des accords de de défense entretenu avec les, les différents pays en fonction aussi de l'actualité liée à la lutte contre le terrorisme et ça évidemment, je répondrai à vos questions. Sur ce point tout à l'heure l'heure 3ème famille évidemment de base, ce sont au fond des positionnements. Qui se font sur le régime des opérations extérieures, notamment aux côtés des forces locales. C'est vrai dans deux immenses pays dont la sécurité évidemment et la stabilité sont clés que sont le Tchad d'une part et le Niger. Le Niger pour l'ensemble des sénateurs qui ont pu s'y rendre. Récemment, je pense que ça incarne ce le mieux en tout cas l'offre française rénovée en matière d'appui au combat, on est véritablement là pour le coup dans une logique où on est aux côtés du partenaire nigérien. Ne fait pas à la place de on ne se substitue pas, on ne le sort et on ne engage un certain nombre de missions que, à la demande justement des autorités nigériennes dans un dialogue à la fois sécuritaire militaire un dialogue politique ah dialogue diplomatique et on commence à voir des résultats tout à fait probant sur le terrain. Je suis frappé de voir notamment sur la région qui Labeyrie dans lequel on avait pratiquement 33% de de de surface agricole exploitable seulement à cause de la présence de groupes terroristes armés désormais en plusieurs mois d'opérations avec les forces militaires françaises et nigériennes nigériennes et françaises. On est passé de 33% de surface. Cultivable à un taux de 65%. Cela dit quelque chose évidemment de l'efficacité des missions qui sont menées dans une forme d'ailleurs de discrétion voire même si j'ai été provoquant à Paris d'indifférence alors que pour le coup, le Niger est engagé dans un con très courageux, c'est le moins que l'on puisse dire contre les groupes armés terroristes et c'est quand même de par le Niger, que nous avons aussi le succès du déménagement des éléments de Barkhane du Mali vers le Niger. Il y a un an et sur l'ensemble de la stabilité dans la zone sahélo-saharienne, donc je pense qu'il, là aussi En saluant les efforts du président Bazoum. Et de, et de son armée. 5ème Point au fond la mise à jour de cette présence militaire française que le président de la République l'a annoncé il y a maintenant plusieurs mois. Elle va se faire sur la base de quelques points de doctrine dont j'aimerais veut clarifier les choses devant la Haute Assemblée. Hein je l'ai dit c'est condition désormais du succès parce qu'il y a cette guerre informationnelle qui est menée par un certain nombre de compétiteurs parce qu'il nous faut aussi apprendre de nos échecs ou en tout cas tirer des leçons sans faire les inspecteurs des travaux finis comme parfois certains voudraient le faire mais en tout cas en regardant lucidement. Ce qui a été la fin de Barkhane, c'est de se dire qu'on ne doit plus se substituer aux États souverains africains dans l'émission de lutte contre le terrorisme. Être présent et répondre à une demande à l'ou un appui oui faire à la place de inévitablement ça nous expose et ça ne donne pas satisfaction à la fin à la mission sur le terrain militaire mais aussi bien sûr sur le terrain diplomatique et sur le terrain. Politique, ça veut dire aussi que désormais il faut aussi que le besoin de France sur le terrain militaire, passe par une expression de volonté en clair ce que l'on ferait entre n'importe quel État souverain d'un État souverain, un autre dans le respect justement de cette souveraineté et en disant au fond qu'est-ce que vous voulez. Et qu'est-ce que nous sommes prêts à faire et si ça fonctionne au Niger ou si ça fonctionne à Djibouti pour prendre ces 2 exemples, là, c'est bel et bien parce qu'il y a beaucoup d'écoute et beaucoup d'attention qui est portée à l'expression du besoin justement des partenaires concernés et ça c'est évidemment un chemin qu'il nous faut prendre aussi sur les autres pays dans lequel nous avons des forces qui est actuellement en cours. Pour le Sénégal pour le Gabon pour ne citer que ces 2 exemples mais aussi pour la RC. La 2ème des choses, il nous faut réfléchir à la taille de nos empreintes militaire. Le temps est passé, nous avons parfois des situations qui sont pas toujours efficientes pour les forces armées prendre un exemple très concret au Sénégal on n'avait pas une base, au fond, mais vous avez pratiquement 7 à 8 empreinte. Militaire française dans l'ensemble de Dakar agglomération ça ne donne pas satisfaction aux forces armées depuis longtemps et de fait on s'aperçoit qu'on a des modules aujourd'hui des des terrains militaires français qui sont ouverts à la formation pour le partenaire sénégalais et dont on aurait beaucoup intérêt à bascule dans une forme de cogestion. de l'intégralité de la base française je vous rassure évidemment mais sur certains éléments dès lors que vous êtes dans un partenariat de formation, vous avez déjà une intimité stratégique qui est très très forte avec le partenaire, vous êtes déjà dans une forme de confiance très abouti, c'est le moins que l'on puisse dire et donc au fond, il nous faut permettre aussi d'être beaucoup plus moderne est beaucoup plus de 9 vendent à la manière de gérer ses empreintes militaire, ça c'est un point qui est clé, sur lequel les choses avancent bien et là aussi si on regarde de près l'ensemble des empreintes, elles ne sont pas comparables les unes aux autres. Les éléments français au Gabon. Au Sénégal, au fond, sont déjà très ouvert sur la ville avec des associations, des crèches, des écoles qui sont parfois en plein milieu du camp militaire là où vous avez par exemple le camp de Port-Bouët à Abidjan, qui est un, une grosse caserne en quelque sorte ce qui est à l'extérieur de la ville et qui donne l'impression d'être très déconnecté de la vie justement. De de la vie ivoirienne du quotidien si j'ose dire, donc là évidemment c'est une réflexion qui est clé tout ça de ceux qu'ont été maire ici. Comparaison n'est pas raison ou élus municipaux en savent quelque chose. On ne peut pas déconnecter désormais une emprise militaire de son environnement environnement civils cette là aussi une des grandes conclusions que nous avons sur ce qui se passe actuellement en Afrique d'autres partenaires et alliés l'ont déjà fait, il n'y a aucune raison que nous prenons du retard en la matière 3ème chose. Il nous faut proposer désormais un catalogue de formation un jour. Je pense que nous avons été parfois trop satisfaits de nous-mêmes pour être clair et de l'offre de formation telle qualité produit soyons bien d'accord. Ce que nous faisions était de qualité mais malheureusement avait tendance à mal vieillir. C'est-à-dire que là où nous apportions des éléments de formation d'autres partenaires ou pays, la Turquie, Israël, pour ne citer que ces deux là parfois l'Algérie commencer à proposer justement des formations sur des segments nouveaux lutte anti-drone ou prise en main de certains drone. Où évidemment culture au initiation au sujet du cyber de la guerre électronique et ça pour le coup, c'est un des éléments qui va me conduire aussi à, à prendre des décisions d'organisations aussi différentes de nos forces prépositionnées plutôt que d'avoir des séjours longs avec des métiers fixe ou statique plutôt aller vers des séjours plus courts avec des compagnies ou des bataillons de militaires français pour pour parfois un mois 2 mois 3 mois parfois aussi composé de réservistes. Je pense que c'est un des points aussi clé avec nous réservistes pour être en situation d'avoir une offre de formation beaucoup plus large. Parfois. Très de masse, si j'ose dire sur des fonctions simples désarmement dit ED protection individuelle combat d'infanterie classique mais aussi parfois sur le haut du spectre sur des sujets avec plus de valeur ajoutée puisque là pour le coup, c'est un des points sur lequel si nous ne prenons pas garde, nous pourrions prendre du retard. Si ce n'est déjà fait pour être honnête, et donc évidemment il nous faut, il nous faut avancer enfin pour avancer dans les éléments de doctrine. Il nous faut réouvrir nos écoles militaires sous-officiers et officiers j'insiste aussi sur sous-officier sur le territoire national. La fin du service militaire. L'avènement de notre armée de métiers qui était une bonne chose par ailleurs. Les différentes diminutions de crédits que le ministère de la défense ou des armées ont pu connaître à travers le temps font que de petit à petit. Saint-Cyr-Coëtquidan école navale Salon de Provence, pour citer les 3 écoles d'officiers mais il y en a d'autres évidemment polytechnique aussi on finit par exclure de plus en plus de stagiaires des pays amis des pays partenaires d'Afrique, là où vous aviez des. Dans les années 80 ou 90, avec parfois plusieurs dizaines de jeunes aspirant, sous lieutenant il suit des armées africaines. On se retrouve aujourd'hui parfois avec un, deux 3 élèves officiers par courtes donc après on peut toujours parler d'influence. Évidemment tout ça a ses limites et donc moi j'ai demandé à ce que nos écoles soient réouvertes. Avec un objectif de 600 stagiaires. Venant des pays d'Afrique chaque année à horizon 2030, avec évidemment une pente pour ce faire, mais qui est un point clé et qui suicident je le crois beaucoup d'adhésion de la part des partenaires que nous avons interrogés en la matière vain une réflexion à avoir sur le capacitaire sur les équipements et sur l'armement. Notre base industrielle et technologique de défense avec toutes les qualités qu'on lui connaît. A pris évidemment de bonnes habitudes à l'exportation d'armes vers les gros contrats pour les grands pays, c'est une bonne chose. On s'en réjouit tous. Force est de constater que les armées des pays partenaires. Sont aussi armées qui accomplissent des efforts budgétaires importants pour monter en puissance l'armée sénégalaise et l'armée ivoirienne n'a rien à voir aujourd'hui avec celle que nous avons pu connaître il y a 10 ou 15 ans. Or les besoins d'équipement en capacitaire sont aussi présents. Et force est de constater et je sais qu'un certain nombre de sénateurs qui ont fait. Quelques voyages récemment l'ont entendu comme moi que parfois nos industriels ont pu on va dire et conduire un certain nombre d'armées de pays amis en disant au fond ce sont des contrats qui sont trop faibles ou dont la quantité n'est pas suffisamment satisfaisantes, D'autres partenaires ou compétiteurs et concurrents ont pris notre place, donc là il y a évidemment une réflexion clé avec la DGA avec la BITD, avec aussi le monde bancaire et avec. BPI et d'autres organismes pour être capable justement d'avoir des solutions pour l'ensemble de ces pays pour leur permettent de continuer à monter en puissance, on revient entre faire avec être aux côtés aider à faire faire. Évidemment, ça passe aussi par les équipements et on ne peut pas ne pas le voir cette aussi une réflexion que j'en termine par là, monsieur le président du Sénat, Mesdames, messieurs les sénateurs. Peut-être aussi pour dire que on y reviendra dans le cas de la discussion de la programmation militaire mais il nous faut aussi renforcer nos réseaux d'attaché de défense. La ministre est revenue sur le le renforcement du réseau diplomatique, ça vaut aussi évidemment pour les attachés de défense pour les attachés d'armement ont figurez-vous que aucune ambassade en Afrique aujourd'hui ne dispose attaché d'armement de de de de la DGA. Ce qui est évidemment là aussi un non-sens. Il nous faut évidemment, remonter en puissance que cela passe évidemment par les capacités expéditionnaires. On l'a vu avec l'opération sagittaire évidemment pour l'évacuation de Khartoum. C'est vrai pour d'autres opérations ça pose la question aussi de la cohérence et de la masse. On y revient là encore avoir beaucoup d'A400M c'est bien avoir des A400M qui vole avec une interopérabilité forces spéciales qui vont avec, je le répéterai encore à Longwy. Mais c'est ce qui nous permet d'y arriver ça pour le coup, on a des des perspectives de contrats opérationnels nouveau, à mon avis en matière expéditionnaire à l'avenir qui nous permettra d'avoir beaucoup plus d'agilité dans notre manière de de d'avancer la question du renseignement sur lequel je mettant pas ici ça a été traité lors de la DPR mais enfin qui étaient évidemment sur un sujet clé, notamment en matière de lutte contre le terrorisme ont conclusion dans les axes d'effort je vous ai beaucoup parlé des pays francophones, au fond, dans lequel nous avions deux bases parce que c'était la commande qui m'avait été donné d'éclairer le Sénat sur la manoeuvre en cours pour les bases. Donc j'ai fait ce parti pris, si j'ose dire. Éditorial dans mon propos que de vous éclairer. Je l'espère complètement sur ce sujet. Il est clair que les sujets de sécurité de défense s'applique aussi à l'Afrique. Lusophone et anglophone. Avec des pays qui sont eux aussi largement confrontée la lutte contre le terrorisme. Je vais citer quand même la question du Mozambique qui nous intéressent très directement et pour cause, on est dans le bouchon du canal du Mozambique. Nous avons l'archipel de Mayotte hein pas de la. L'Angola dans lequel le président de la République s'est rendu il y a peu de temps. Voilà ce ne veux pas tous les citer, mais d'autres pays dans lequel nous n'avons pas de force mais pour autant, nous avons des perspectives d'accord de défense potentiel à renouveler ou à raffermir en matière de partenariat là aussi en matière de capacitaire. Je rappelle quand même à la Haute Assemblée, que nous avons signé un contrat pour une offre satellitaire avec. En En matière de renseignement avec l'Angola. Ce qui n'est pas forcément intuitifs de prime abord, mais qui montre bien là aussi que si on est compétitifs on est capables aussi d'aider les partenaires sur des segments technologiques nouveaux. Dernier point, il y a quand même un esprit de Takuba. Qui demeurent encore parmi les partenaires européens. Parfois, les questions de l'Europe de la défense mérite d'être traité avec beaucoup de précaution, il faut reconnaître que pour le coup, nous sommes en dehors de l'OTAN. Nous sommes en dehors des des des cercles classiques d'intervention et que la France a su est l'armée française par ses compétences, a su emmener. Beaucoup de partenaires européens en matière expéditionnaire et que pour le coup, beaucoup de pays d'Europe ont compris l'intérêt aussi de de d'aider les pays d'Afrique à lutter contre le terrorisme cet esprit de Takuba, pour le coup, il faut qu'on arrive à le faire vivre, parce que c'est une véritable avancée. Voilà. Mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le président du Sénat, monsieur le président de la commission, ce que je voulais évoquer devant la Haute Assemblée sur l'articulation de la présence française en Afrique. Je vous remercie. Merci monsieur Mounier. La parole est maintenant aux orateurs des groupes tout d'abord le président Christian Cambon pour le groupe Les Républicains. Monsieur Monsieur le Président Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Au cours des 60 dernières années. La relation que nous entretenons avec les pays africains à rythmé comme nul autre. La vie de notre pays de sa diplomatie de sa coopération et de ses armées. Cette histoire est le reflet d'une longue histoire commune. Une histoire qui porte ses indéniables part d'ombre auquel il faut savoir se confronter mais une histoire qui fut aussi brillante d'engagement sincère d'amitié profonde et de réalisation admirable. Cette relation si singulière chaque président de la République a voulu lui imprimer sa marque, lui donner un nouvel élan, une nouvelle perspective ou une nouvelle méthode. L'actuel chef de l'État ne fait pas exception à cette règle. Lui qui, en policier lui qui ambitionnait en 2017 à Ouagadougou d'écrire, je cite, une nouvelle relation d'amitié avec le continent africain. Et pourtant nous voilà en 2023, confronté à cette question qui s'impose chaque jour avec davantage de force. La France et l'Afrique partagent un passé mais partage-t-elle encore un avenir. Le coeur presque autant que la raison m'incite bien sûr à ils répondent sans ambages par l'affirmative. Mais le fait même de formule et cette interrogation impose de procéder à un constat lucide et sans concession de la situation. Bien sûr et vous l'avez rappelé, la France reste sur le continent africain, un acteur clé dans un grand nombre de domaines. Mais depuis 20 ans. Sa présence et son influence s'ils font de plus en plus relative. Dans ce laps de temps. Ses parts de marché ont fondu de moitié depuis 2007. La Chine a remplacé la France comme premier exportateur vers le continent africain. Depuis 2017, elle a perdu son statut de 1er fournisseur européen au profit de l'Allemagne et depuis l'année dernière, elle n'est même plus le 1er partenaire commercial d'aucun des pays du Maghreb. Les épisodes de tension se sont multipliées en Afrique subsaharienne, mais aussi en Afrique du Nord ou le principal résultat du rapprochement tenté avec l'Algérie et pour l'heure une prise distance une prise de distance de notre allié marocain. Le rayonnement de la culture française s'estompe également. En 2018 59 % des 300 millions de locuteurs français dans le monde était africain pourtant des pays francophones comme le Rwanda le Togo ou le Gabon. On fait le choix de rejoint le Commonwealth, voire pour certains d'adopter l'anglais comme langue officielle ou comme langue d'enseignement, le Maroc et l'Algérie envisageraient même de s'engager dans une voie similaire. Et si la France reste le 1er pays de destination des étudiants africains. Vous l'avez dit Madame la Ministre cette capacité à attirer les futures élites du continent pour les former et malheureusement en Net recul par rapport à d'autres destinations. Mais surtout, nous devons faire face. Dorénavant au mur de ce que l'on appelle communément le sentiment anti-français. Certes, nous pourrions être tentés de le relativiser de n'y voir qu'a un effet de loupe créée par quelques milliers d'activistes ou de des informateurs aux motivations douteuses. Ce serait une erreur, ce serait une erreur car le phénomène est devenu incontournable. Il a joué un rôle majeur dans le départ contraint de nos armées au Mali, au Burkina Faso ou en République centrafricaine. Le constat est cruel. Malgré l'engagement remarquable de nos militaires contre le terrorisme islamiste et le sacrifice de 53 d'entre eux dont le souvenir est présente dans notre coeur à tous jamais la France n'a été dans ces pays comme d'autres. Tant critiqué et parfois rejeté. ce ressentiment plonge bien sûr ses racines dans la colonisation ou dans certains errements de la période post-coloniale. Mais il tient aussi au fait que tout simplement l'Afrique a profondément changé. Il y avait 275 millions d'Africains. En 1960, ils sont aujourd'hui 1 milliard 200 millions dont plus de la moitié a moins de 25 ans, une véritable bascule générationnelle s'est opéré distants dans nos Liens diplomatiques, militaires et culturel. Les nouvelles générations, les nouvelles élites africaines au coeur de l'école de l'essor économique du continent sont aussi celles de la globalisation. Le monde désormais se pressent à la porte de l'Afrique, les pays africains et c'est bien normal multiplie les partenariats, loin de toute relation exclusive cette réalité et les attentes qui en découlent concernant la relation avec la France. Sans doute ne les avons-nous pas suffisamment observé ni même intégré. Ne soyons pas non plus naïf. Certains de nos compétiteurs stratégique font tout pour nous évincer et cherche pour cela accroître le sentiment anti- français dans ce domaine. L'affaire du prétendu charnier de Gossi nous a une nouvelle fois montré que tous les coups contre la France était permis. Alors. Comment réagir à cette nouvelle donne naturellement nous devons entendre les reproches qui nous sont faits les plus. Comme les plus injustes et y répondre par les mots, mais aussi par les actes. cela ne signifie en aucun cas que nous devions les intériorisé au point qu'il guide à chaque instant notre attitude vis à vis de l'Afrique et des Africains. Comment en effet présenter une image attractive de notre pays si finalement nous acceptons à notre for intérieur qu'elles soient dévalorisés alors refusant le discours de ci, de ceux qui dans le passé ne voudrait voir qu'un passif Nando sont pas à la rhétorique de ceux qui mettent la France en accusation permanente et pour qui elle aura toujours tort quoi elle dise ou quoi qu'elle fasse. Assumons par ailleurs franchement la promotion de nos intérêts. Car oui, la France a des intérêts en Afrique comme certains voudraient le faire croire, dans une domination économique fantasmer à travers du franc CFA ou dans une exploitation supposément prédatrice des ressources minières nos véritables intérêts mes chers collègues sont bien ailleurs sur le plan sécuritaire. Nous avons intérêt à ce qu'il y ait moins de crises sur le continent car tout conflit peut générer des effets négatifs de l'autre côté de la Méditerranée de la prolifération des armes au terrorisme en passant bien sûr par l'immigration irrégulière. Sur le plan des équilibres internationaux. Nous souhaitons nous fonder sur nos Liens anciens avec certains pays africains pour continuer à appuyer mutuellement nos positions au sein des instances internationales. Sur le plan économique, enfin. Il est évident que, comme le reste du monde. Nous avons intérêt à ce que l'Afrique continue de s'affirmer comme un relais d'innovation et de prospérité. Mais pour oeuvrer efficacement sur tous ces plans. Il nous faut avant tout restaurer les moyens de notre influence. La revue nationale stratégique de novembre 2022 a justement fait de cette dimension. Une nouvelle fonction stratégique. Si je voulais faire de l'ironie. Je dirais qu'il était temps de redécouvrir que la diplomatie consiste à avoir de l'influence plus sérieusement la cohérence de notre action dans ce domaine interroge parfois tant le hiatus est important entre des habitudes des ambitions affichées et le sort que nous réservons parfois à notre propre diplomatie. Avec une réforme qui nie parfois ses spécificités et son savoir-faire et des moyens qui ont été drastiquement réduit depuis 30 ans. La situation est inquiétante, même si Madame. Je souhaite vous donnez Madame la Ministre acte du fait que vous avez stopper cette hémorragie. Et je souhaite le reconnaître ici. Combien d'agents malgré tout sont aujourd'hui affectés à la veille et à la diffusion d'informations au au sein de chacun de nos postes diplomatiques dans les pays d'Afrique de l'Ouest une poignée parfois seulement un stagiaire. Services de coopération et d'actions culturelles, quant à eux se réduisent, année après année. À contrario, les crédits consacrés à l'aide au développement ont beaucoup commenté, c'est très bien, c'est non seulement conforme aux engagements internationaux de la France, mais c'est surtout essentiel. Permettez-moi Madame la Ministre de profiter de cette intervention pour regretter que malgré nos appels répétés, la commission d'évaluation des politiques de de soutien au développement prévu par une loi d'orientation du 4 août 2021 n'est toujours pas entamé ses travaux et du reste ne soit toujours pas constituent. Quand elle le fera cette commission elle constatera sans doute qu'il est indispensable de recentrer notre politique de solidarité internationale sur quelques priorités fondamentales que nous martelant en commission nourrir soigner voilà les domaines où notre aide et la plus attendue là où elle peut porter ses meilleurs fruits bien sûr notre action peut et elle doit être conduite dans le respect du climat et de la bonne gouvernance. Mais c'est bien sûr ses dimensions vital pour les populations qu'elle aura le plus de Trop longtemps notre aide au développement à fonctionner en vase clos, sans voir que nos partenaires eux font proche d'une approche beaucoup plus intégrés notre assistance technique formidable levier d'influence et d'exportation de notre savoir-faire par le passé est devenue extrêmement réduite. Par comparaison l'organisme allemand. Là j'ai Réalise un chiffre d'affaires de 3 milliards 700 millions d'euros et emploie 23.600 personnes expertes iFrance. 339 millions d'euros. 1400 personnes. Il faut en outre reprendre le contrôle de notre aide multilatérale à l'Afrique. Plus de la moitié des contributions du Royaume-Uni. Plus du tiers des contributions allemande aux organismes multilatéraux sont fléchés vers leurs propres priorités d'action pour nous ce n'est que 1%. Quelle perte d'influence par rapport à nos partenaires. Il faut aussi compléter cette approche en incitant et en accompagnant bien davantage nos entreprises. Vous l'avez dit Madame la Ministre à s'implanter à investir à commercer avec le continent car c'est aussi comme cela qui sont bien souvent préoccupations qui sont bien souvent d'ordre économique. Enfin, reste la question centrale structurante de notre coopération militaire. Une opération telle que Barkhane malgré ses succès indéniable et j'approuve tout à fait ce que vous avez eu l'occasion de dire, Monsieur le Ministre, sur ce sujet. Cette opération constitue sans doute peut être une anomalie par sa durée particulièrement longue faute de progrès sur la solution politique. La France s'est retrouvé exposé en première ligne pendant des années vulnérables face à la propagande et russes de Wagner et de tous ceux qui ont intérêt à notre départ. Pourtant, cette opération a aussi enclencher des partenariats utiles ainsi au Niger nos forces collabore efficacement sous commandement nigérien à la lutte contre les groupes terroristes ces coopérations doivent être poursuivis car elles permettent à nos partenaires de monter en puissance. Dans son discours de février dernier, le président de la République a proposé de les inscrire dans le cadre d'un nouveau partenariat sécuritaire. Certains axes dégagés à cette occasion nous semble de bon sens ainsi. Moi je partage la volonté de mieux répondre aux demandes ponctuelles de nos partenaires. Je pense par exemple à l'appui aux renseignements où nous pouvons apporter notre connaissance et notre capacité de surveillance des groupes djihadistes qui tentent de s'infiltrer dans le nord de la Côte d'Ivoire du Bénin ou du Togo. Je souscris aussi au constat selon lequel nous ne vaincront pas les terroristes à la place des pays concernés tout appui opérationnel. Il doit donc dorénavant rester ponctuelles discret et efficace. Mais s'agissant de nos bases militaires. Monsieur le Ministre, vous connaissez ma position est celle de la commission. C'est bah sont essentiels et la récente opération sagittaire brillamment conduite à partir de Djibouti pour évacuer nos ressortissants présents au Soudan en est une nouvelle preuve. Nos compétiteurs stratégiques sont d'ailleurs ceux-là mêmes qui ont convaincu de cette importance et notamment la Chine qui a pressé de Djibouti cherche à ouvrir une base dans le Golfe de Guinée. Je ne suis pas hostile à ce que nous travaillons d'une manière différente, en cherchant à tenir compte du contexte local de chaque base pour mieux nous y adapter. Mais s'agissant d'un outil militaire je souhaite souligner que ses bases sont aussi l'expression de notre souveraineté qui par définition ne se partage pas, naturellement, il appartient en contrepartie aux États. Et à eux seuls de décider s'ils Acted. Ou non notre notre présence Mais l'annonce de leur co-gestion me pose un problème au plan conceptuel il m'en posant aussi au plan opérationnel, car dans ce cadre. Serions-nous toujours capables demain de lancer dans l'urgence une opération telle que sagittaire. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, nous sommes à un moment charnière de notre relation avec le continent africain et ce débat avait pour but de vous donner l'occasion de préciser vos priorités. Soyons objectif, rien n'est plus acquis dans ce nouvel environnement ultraconcurrentiel. Où de nombreux pays y compris nos partenaires européens du reste tentent de gagner de nouvelles positions en Afrique, notre pays s'il veut continuer à jouer un rôle de 1er plan devra tirer les leçons parfois douloureuse de ces 20 dernières années et de ces quelques échecs sur tous les plans, nous devrons nous adapter nous battre nous remettre en question parfois mais aussi savoir se montrer fier de ce que la France a accompli en Afrique. La palette des outils à notre disposition et large. Il faut désormais les mettre en cohérence autour du cap clair et cohérent qui leur fait encore défaut avec un seul mot d'ordre, parions sur l'Afrique et parions sur la France, je vous remercie. La parole est à notre collègue Marie-Arlette Carlotti pour le groupe social. Écologiste et républicain. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président Cambon, mes chers collègues. Ce débat sur la politique de la France en Afrique. Le groupe socialiste la souhaiter mais dans une forme autre que ça fait change extrêmement formelle qui ne nous permet pas vraiment d'exercer pleinement notre rôle de parlementaire. Il intervient dans un contexte particulièrement douloureux, celui du déclin relatif de l'influence de la France sur le continent africain, marqué par le rejet spectaculaire de la présence militaire au Mali et au Burkina Faso. Pour beaucoup, ça a été un révélateur. Nous savons que les choses remonte à bien plus longtemps. Alors que dans les années 90, le continent était abandonné, il est désormais courtisé par de nombreux pays la Russie bien sûr mais aussi la Chine et depuis bien longtemps, les États-Unis, le Japon, la Turquie, les Émirats arabes unis. Tous ont développé un appétit à l'égard de l'Afrique tout son nom compétiteurs. Nous avons perdu nos Liens privilégiés exclusif avec les États africains. que nos relations deviennent ordinaires, et ne soient plus marquée du sceau de la singularité. Alors que la hiérarchie du monde change l'Afrique veut être considéré comme un acteur de plein droit sur la scène internationale. C'est un défi géopolitique majeur que le président Macron a pointé du doigt et qu'il convient de traduire dans les faits. Au fil des ans, la société civile africaine a changé la jeunesse qui n'a pas connu les combats pour l'indépendance trouve dans un sentiment anti-coloniale le chemin alternatif vers l'émancipation une partie c'est même fortement radicalisés le panafricanisme s'est développée, partisan d'une rupture franche avec l'Occident vieillissant qui continue pourtant à vouloir imposer son ordre mondial ce conflit avec l'Ouest permet permet d'ailleurs de réhabiliter les groupes djihadistes auprès des populations et la Russie. Il fait son miel. L'Afrique prend ses distances avec la France qui a perdu sa position privilégiée mais pourquoi l'aurait-elle parce que elle ne se distingue pas elle ne développe pas une diplomatie original des Liens nouveaux équilibré et respectueux. Certes le président proclame la fin de la Françafrique. Bon ça concerne que l'Afrique francophone hein. Mais ce n'est pas nouveau depuis Georges Pompidou tous ses prédécesseurs l'ont fait avant lui et pourtant et pourtant nous avons continué à surfer sur nos relations anciennes basée sur notre histoire coloniale emprunte de corruption et de clientélisme, de double langage et d'arrogance. Du fait de l'importance du continent africain et de son affirmation sur la scène internationale, la France ne peut se passer d'une politique à l'égard de l'Afrique. Mais elle doit changer d'approche. Le 27 février. Emmanuel Macron a prononcé un discours qui se voulait fondateur. Nous attendions qu'il clarifie donc les nouvelles orientations de sa politique dans un contexte pour le moins tendues. Au lieu de ça, cette intervention s'inscrit plutôt dans la continuité et sur beaucoup de points restent floues. En tout état de cause, elle ne constitue pas les prémices d'une nouvelle politique africaine sur le plan militaire. Je tiens à rendre hommage à l'engagement de nos soldats lors des opérations Serval et Barkhane et vous avez raison, Monsieur le Ministre, nous avons eu, ils ont eu de vrai succès

franchement on ne peut pas dire que ce soit une vraie réussite. En tout cas je ne le vois pas comme une réussite. Je trouve que l'Union européenne a montré de ce point de vue sa faiblesse. Or, si elle veut être. Si elle ne veut pas être la grande perdante de la compétition qui s'est engagée et en Méditerranée et sur le continent. Elle doit s'à s'impliquer davantage dans cette zone instable en considérant l'Afrique ni comme un libre-service une réserve de richesse et de matières premières rares ni comme une menace vis-à-vis de laquelle il faudrait se barricader. Nous ne sommes plus le gendarme de l'Afrique, vous l'avez dit, ce temps est révolu. Alors il nous faut changer de modèle. Le président de la République encore là, a affirmé l'influence de la France de se mesurera plus au nombre de nos opérations militaires ni aux nombres de nos bases il préconise la réduction de l'empreinte directe de nos forces au profit d'un soutien aux forces de sécurité de la région. Vous avez développé beaucoup de choses. Monsieur le Ministre tout à l'heure alors. Cela signifie-t-il que nous entrons dans une phase de repli ou est-ce que nous allons continuer à nous mobiliser contre le djihadisme qui touche désormais des pays qui jusqu'alors on était prémuni comme le Mozambique. Dans le domaine de l'aide au développement. Emmanuel Macron a fait des annonces aussi lors de l'Élysée sur le fond, nous avons bien entendu que la notion d'aide au développement est à proscrire. Selon un proverbe africain. La main qui donne est au dessus de celle qui reçoit. Ils nous invitent à passer d'une logique de l'aide à une logique d'investissement solidaire et partenariale, là aussi franchement ça s'inscrit dans une rhétorique déjà ancienne et malheureusement les Africains ont l'habitude de ces déclarations non suivies d'effet, si les annonces présidentielles confirme la mobilisation de la France en faveur de la solidarité internationale notamment droits humains climat santé éducation jeunesse égalité femme-homme nous regrettons cependant que l'eau et l'assainissement n'ait pas été cité lorsque alors qu'ils étaient une priorité sectorielles que nous avons inscrit dans la loi du 4 août 2021. Mais ce sont les organisations de la société civile qui ont été les grandes oubliées des priorités. Proposées par le président. Les ONG françaises bien sûr mais aussi les ONG des pays partenaires par leur proximité et leur engagement auprès des populations, elle joue un rôle majeur. Nous devons en faire des partenaires privilégiés de notre politique. Si les rappeler dans le discours du président, les efforts financiers engagés par la France jusqu'en 2022, la trajectoire des financements a cependant été éludé les engagements de la France sont pourtant clairs sur ce sujet ils sont inscrits dans la loi du 4 août 2021 qui a affiche une trajectoire visant à louer 07% de revenu national national brut de la France à l'aide publique au développement, à l'horizon 2025. Nous sommes absolument opposés à rouvrir un débat qui a déjà été tranchée et nous souhaitons que cette trajectoire soit maintenu. En fait, il nous manque toujours cet outil d'évaluation de nos politiques publiques d'aide au développement prévu par la loi. Voilà 2 ans, 2 ans, que la commission d'évaluation aurait dû être mis en place. Pourquoi tant de tergiversations. Nous vous rappelons que nous avons adopté au Sénat le rattachement de la commission auprès de la Cour des comptes. Dans la stratégie 3D que le gouvernement a théorisé que je trouve qu'il n'a pas réussi non plus l'appareil militaire de défense et de développement était étroitement liée à la diplomatie. Sur ce point, une question se pose. La diplomatie française fait-elle preuve de naïveté ou d'aveuglement, avons-nous sous-estimé la puissance du ressentiment et de la rancune que ces pays nourrissait à l'égard de la France. Surtout si l'histoire était convoqué par une propagande hostile et je ne le nie pas, au contraire. Mais moi je ne le crois pas, je pense plutôt que notre logiciel politico-diplomatique est ancien et obsolète. On fait de la diplomatie comme on en faisait il y a encore quelques décennies. À l'époque où la France faisait et défaisait les régimes en place qu'elle en avait les moyens financiers et humains. La France a oublié, peut être que l'Afrique des gouvernants c'est pas forcément celle des peuples. Depuis quelques années les moyens donnés à la diplomatie française sont trop faibles comparés à ceux des autres pays et même si l'Afrique n'est pas la plus mal lotie n'est pas plus démunis que d'autres pays, nos petites ambassades sont contraintes de fonctionner en couteau suisse ainsi au Sahel, la présence de la France a été beaucoup plus militaire que diplomatique et la réforme d'Emmanuel Macron du corps diplomatique, paru le 16 avril n'a pas apaiser nos inquiétudes, elle n'apporte aucune amélioration n'Ukrainian même au contraire qu'elle fragilise l'appareil diplomatique français, ce qui serait affaiblir le rayonnement de la France c'est une donc une situation inquiétante au moment où nous avons vraiment besoin de diplomate aguerri aguerri et. Je veux d'ailleurs leur rendre hommage, le président de la République a essayé d'ouvrir d'autres voies de dialogue lors du sommet Afrique-France à Montpellier j'y été. Ce fut un très bel événement mais qu'en reste-t-il un observatoire pour la démocratie. À quoi sert cette initiative. La démocratie ne se décrète pas en laboratoire, elle est portée par un mouvement populaire. Elle est le fruit d'un engagement politique. Emmanuel Macron a voulu une démarche moderniste. Il a proposé un schéma surannée et à contresens et de la même manière. Alors que le franc CFA fait l'objet de débats passionnés depuis des décennies. Une annonce venue d'en haut, entre le président Ouattara et le président Macron sans processus de décision auprès des autres chefs d'État sans consulter. Bien entendu, les populations ne peut que faire débat. Une décision imposée et d'une décision suspecte toujours à quoi sert donc de vouloir imposer nos modèles clés en main, il suffit de soutenir une gouvernance respectueuse des droits humains sans imposer un agenda démocratique irréaliste. Le chef d'État a insisté sur la démocratie, la liberté dans son discours du 27 février à l'Élysée. Or, depuis son élection il s'est certes très souvent rendu en Afrique mais souvent dans les pays les moins démocratiques du continent et qui abrite les ancien autocrate. Les plus anciens autocrate ainsi que leur dynastie. Il semble que la réelle politique le dépasse toujours et nous nous reprochons pas d'ailleurs à Emmanuel Macron de pratiquer la réelle politique afin de croire de faire progresser l'influence de la France. Nous mesurons combien l'exercice est difficile, ce que nous condamnons, c'est le double langage, on accepte le pouvoir militaire au Tchad et on le condamne au Mali. Nous perdons toute crédibilité lorsque nous défendons des valeurs à géométrie variable. Nous devons nous montrer plus attentifs aussi aux tragédie qui touche le continent les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité en Éthiopie au Soudan en RDC de stratégies en raison de de de tragédie en raison du réchauffement climatique elle frappait déjà les les régions de la Corne de l'Afrique, la situation s'est aggravée, nous le savons par la non livraison de céréales à bas prix venue de l'Europe de l'Est sans que et on est en train peut-être d'y remédier sans que ni l'Union européenne et la France ne puisse en prendre le relais de façon claire, précise, du moins à court terme pour faire face à la disette. En République Centrafrique et au Burkina Faso, vous le, vous le savez le chantage alimentaire constitue un des facteurs déterminants de la montée de l'influence de la Russie. Ces crises alimentaires vont immanquablement déboucher vers une nouvelle crise migratoire. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, sachez que lors du débat sur l'immigration. Nous veillerons à ce que notre politique de développement ne soient pas assujettis aux enjeux de politique intérieure et dites à monsieur au ministre Darmanin que sa politique restrictive des visas à couper les Liens indéfectibles avec les Africains et particulièrement avec la jeunesse. La politique de la France en Afrique est illisible. Elle est blessante blessante car chaque fois que la France exprime elle fait preuve d'un certain paternalisme et de condescendance de maladresse et de propos déplacés qui alimente le sentiment anti-français. Tant auprès des gouvernants que des populations fatigué par ses remarques désobligeantes, les maladresses se multiplient et les incompréhensions demeurent. Nous avons pourtant un formidable atout. Vous en parliez tout à l'heure Madame la Ministre mais nous l'avons pas utiliser quelles que soient les gouvernements, il s'agit de l'espace francophone qui va pouvoir être un vrai vecteur pour nous. En conclusion, il est temps de procéder à des évolutions dans notre dialogue avec l'Afrique, plus exactement bien sûr avec les Afrique mais moi je me suis penché effectivement comme vous Monsieur le Ministre sur l'Afrique francophone, car c'est là que nous avons un lourd héritage à purger. C'est là que nous avons un lourd héritage à purger, faute de quoi le continent entier risque de glisser vers une forme de chaos. Et si la Russie et la Chine qui en tireront immanquablement les bénéfices Eni pillant d'ailleurs l'ensemble des ressources. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Olivier Cadic. Pour le groupe de l'Union centriste.

Monsieur le président du Sénat Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour comprendre l'Afrique. Encore faut-il la connaître. Je m'y suis rendu 57 fois depuis 2015 et elle m'étonne à chaque fois. Je vous livre 3 anecdote. Tout d'abord celle de cet entrepreneur français qui a subi un vol dans sa société. Il se rend à la police, on le renvoie vers la dame au ballet qui lui communique un non après avoir utilisé de ballet croisé après vérification sur sa vidéo surveillance ils découvrent qu'elle a raison. Que dire de ce compatriote qui croit son portefeuille volé à son domicile affolée une personne à son service part précipitamment chez le marabout qui lui révèle que le portefeuille était la vue de tous et que personne ne le voit elle rentre avec le message du marabout le portefeuille et retrouver une heure plus tard. Près de la piscine. Ou encore ce consul général qui fait venir chaque année un coupeur de pluie pour s'assurer de célébrer le 14 juillet au sec. Après 2h de réception le coupeur de pluie lui demande s'il peut partir dès son départ, la pluie se remet à tomber sur le consulat. Les esprits cartésiens seront dubitatif. Notre consul général ne se fait pas rembourser la prestation par le Quai d'Orsay. Olivier le lustre conseillers des Français de l'étranger établies depuis 20 ans en Afrique m'a confié qu'il se refuse à expliquer l'Afrique à quelqu'un qu'il n'y a pas vécu déjà au moins 5 ans. On aborde souvent à tort la stratégie française en Afrique. Par un seul prisme. C'est une erreur car il n'y a pas une Afrique mais des Afrique. Chacune à des problématiques bien distinctes. Même si certaines se recoupent. Emmanuel Macron a visité 25 pays africains depuis sa première élection en mai 2017. Ce qui fait de lui le dirigeant ayant le plus d'engagement diplomatique avec les nations africaines. Pourtant sur le continent africain et plus particulièrement en Afrique de l'ouest et au Sahel. On nous répète que le sentiment anti-français ne cesse de croître. Et si c'était une fête News entretenu illustrant la guerre hybride livrée à la France, pour nous affaiblir. Nous nous fions trop aux réseaux sociaux animée par les activistes. Aujourd'hui, les gens les plus crédibles pour la population sont ceux qui parlent le plus. Pas ce qu'ils disent la vérité. Le mea culpa permanent sur notre passé dans lesquels des soi-disant experts se répandent est ressenti comme une faiblesse sur ce continent. Des grandes entreprises françaises sont l'objet de violentes attaques de la part de représentants d'ONG soutenue par leurs concurrents. Nous avons peut-être perdu une bataille dans la guerre informationnelle l'an dernier au sel. Mais nous n'avons pas perdu la guerre. Vous avez eu raison. Monsieur le Ministre, les militaires de l'opération Barkhane ont été irréprochable. Ils sont notre fierté. Anti-français les Africains. Alors expliquez-moi pourquoi, les chiffres de demandes d'inscriptions pour étudier en France battent des records en Afrique. L'Algérie, on est à 53.000. Elle dépasse pour la première fois le nombre de Marocains d'environ qui est d'environ 30.000 au Togo, après une hausse de 73% sur la période 2016 2021 68 % en 2022 près de 40% d'augmentation déjà enregistré cette année. Un ministre togolais m'a confié que les togolais de France renvoyé plus d'argent Togo que l'aide au développement que nous leurs apportons. Pourquoi donc se détourneraient-ils de nous. Dans beaucoup de pays, il m'a été dit, je ressens une envie de France. Un camerounais m'a dit ce week-end lorsque nous avons le partage de la langue, la proximité plus fortes dans notre inconscient. La France est la plus proche les Liens sont forts. Nos compatriotes installés en Afrique m'ont tous assuré qu'il ne se sent pas menacé en tant que Français. Par contre il est vrai que nous sommes confrontés à une guerre hybride menée contre l'influence de la France et ses intérêts économiques. Avec quelques euros on paye un journalier, aussi bien pour travailler que pour manifester avec un drapeau russe devant l'ambassade de France le sentiment antipolitique française tout comme le sentiment anti- intérêts français n'est pas seulement alimenté par les puissances étrangères et ces proxy dans plusieurs pays des personnes surfent sur du néo-nationalisme font de la France le bouc émissaire de leurs difficultés pour s'imposer politiquement. La collègue Carlotti a parlé des apôtres du panafricanisme, allez voir qui sont derrière. Ces mouvements populistes gagnent en visibilité lorsqu'il s'impose, il se jette dans les bras de la Russie de la Chine de l'Iran et consorts. On le voit au Burkina Faso et au Mali, il trouve un écho auprès des acteurs économiques locaux. Qui en profite pour faire du dégagisme de nos entreprises et participer ainsi à la prédation de leurs activités. Récemment, la filiale des brasseries Castel a été attaqué à coups de cocktails Molotov, en Afrique on suspecte Wagner de nouvelles menaces planent sur cet industriel français emblématique en Afrique qui a fait de la responsabilité sociale de l'entreprise, une marque de fabrique qui fait honneur à notre pays. Monsieur le Ministre, avec l'annonce de retrait de troupes françaises sur le continent. Comment allez-vous défendre nos intérêts économiques et nos entreprises quand ils sont directement attaqués. Comment justifiez-vous ce retrait quand on observe une militarisation accrue de la Chine pour consolider ses Liens diplomatiques et commerciaux avec le continent. Le retrait de Barkhane a fait les affaires des groupes terroristes au Sahel et beaucoup se rendent compte dans les pays avoisinants en voyant la menace progresser. 93%. Des ressources algériennes proviennent du sud algérien. Pour la première fois depuis 17 ans le chef d'État-Major algérien s'est rendu en France comment, analyse-t-il. La situation sécuritaire au Sahel et envisage-t-il une coopération militaire. Le terrorisme islamiste en Afrique le visage du Crime international organisé, structuré, à l'image des gangs criminels que j'ai observé en Amérique latine. Il se drape dans un militantisme religieux pour légitimer les recrutements. Pour lutter contre les gangs au Brésil des milices ont été. Pour protéger des quartiers les il y a les habitants doivent alors se plier aux règles de la milice échangent leur liberté pour obtenir de la sécurité en Afrique, certains pays font appel à la milice Wagner qui se payent sur les ressources du pays, à l'image d'une milice mafieuses, contrairement à ce que certains prétendent, la France n'abandonne pas l'Afrique il y a six mois, j'ai visité l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, près d'Abidjan. Ce centre d'excellence et destinée à appuyer les pays d'Afrique dans la lutte contre le terrorisme. Le modèle de gouvernance de l'Académie franco-ivoirienne est un exemple pour la nouvelle posture de la France en Afrique. Je veux saluer la réunion le 11 mai du 1er conseil d'administration internationale avec les australiens, canadiens Pays-Bas américain. Ce modèle interministérielle porté par l'Académie est un exemple nécessaire en Afrique, il est évident que l'anti-terrorisme soit porté uniquement par l'armée, avec les risques de dérapage sur les populations civiles. Notre modèle est innovant et mérite d'être mieux connue. Combien de pays africains se sont déclarés intéressés par cette initiative. Madame la Ministre, l'attribution, la gestion de l'attribution des visas pour la France est une cause de frustration observée dans de nombreux pays africains. Cela conduit à des décisions défavorables à la France par exemple, certaines entreprises ont préféré se fournir en matériel venant d'un autre pays que la France, de peur de se faire refuser des visas pour une entrée sur le territoire français et risquer de ne pas pouvoir former leur personnel, de manière satisfaisante. Quelles décisions sont prises pour améliorer notre politique d'attribution de visas perçu parfois comme vexatoire en matière d'aide à l'Afrique, il apparaît fondamental d'été, les pays de ce continent à s'organiser dans le domaine de la santé pour faire face à la pénurie de sang il est acheté auprès de donneurs contaminés hépatique, il est une utilisable à 60%. Concernant les médicaments afin de lutter contre les produits contrefaits et aider les industriels à servir le continent. Pourriez-vous porter l'idée de la création d'une agence africaine du médicament. La France porte les valeurs des mots-clés pratique. J'ai personnellement été attristé du renversement du président Roch Kaboré. Un an après sa réélection sans intervenir pour protéger cette démocratie. Le Somaliland est un état du de la Corne de l'Afrique qui a déclaré son indépendance en 91 à l'issue de la guerre civile avec la Somalie, pays actuellement en proie à des conflits depuis plus de 30 ans et qui a des Liens revendiqué avec la Russie, comme en atteste la visite récent du mise malien des Affaires étrangères à Moscou depuis son indépendance, le Somaliland a su garantir une stabilité politique et des élections de président au suffrage universel et de de chambres 5 présidents se sont succédé à la tête du pays depuis son indépendance, allons-nous évoluer sur la question d'une prise en compte officiel du Somaliland pour favoriser son développement où allons-nous continuer à nous limiter aux relations avec Mogadiscio. La France, comme nos partenaires africains ont besoin d'une ligne claire fondée sur le respect mutuel. Cessons de chercher à nous faire aimer. Concentrons-nous sur nos intérêts en faisant valoir nos atouts pour nous faire désirer. Un membre du Parlement togolais l'honorable Ali puis la résumer ainsi hier devant moi à Lomé. Plutôt que plus de France opter pour mieux de France. Je vous remercie. Thierry. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires étrangères et de la défense. Mes chers collègues. Aucune relation internationale n'est aussi complexe ni aussi importante pour l'avenir de notre pays et de notre continent. La politique étrangère de la France en Afrique se trouve à la croisée des chemins, oscillant entre les promesses d'une coopération fructueuse et les traces tenaces de son passé néo- coloniale comme le disait Albert Camus l'amitié n'exigent en rien rien en échange elle grandit librement dans le terreau des valeurs communes. Notre groupe RDPI ce fils licite des résultats de la récente tournée du président de la République en Afrique durant laquelle il s'est rendu au Gabon en Angola. Ainsi qu'en République démocratique du Congo ou et au Congo Brazzaville fin février et début mars. Qui a été marquée par des déclarations importantes et des actions concrètes de la part de notre pays. À titre d'illustration, les programmes de développement durable, les actions en faveur de la gouvernance démocratique et les efforts pour soutenir l'autonomie africaine témoigne d'un désir de réinventer notre relation. Lors de son discours, le président de la République a donc a déclaré au Gabon et affirmé que l'air de la France Afrique était révolu. Cette déclaration reflète la volonté de la France de rompre avec certaines pratiques du passé et de promouvoir un partenariat équilibré et transparent avec les pays africains, un vrai tournant dans cette relation. Après ce tour d'horizon de nos valeurs. Il faut souligner les principaux défis que les pays africains doivent relever d'abord l'environnement. Nous appuyons les mesures prises pour protéger les forêts tropicales et primaire en Afrique protection pour laquelle la France a investi 100 millions d'euros lors du sommet des forêts à Libreville, le 2 mars dernier, Emmanuel Macron a rappelé les engagements pris pris lors de la COP 15 à Montréal et la COP26 à Glasgow pour inverser la déforestation et protéger 30% de la nature. D'ici 2030. Ce format de sommet pourrait être annuel désormais soyons attentifs à la signature d'un nouveau pacte financier CIG Nord lors des travaux prévus à Paris ce mois-ci et au lancement de certificat de biodiversité d'ici la fin de l'année avant la COP 28 à Dubaï, où les premiers contrats. Pays pour la conservation positive pourrait être signé. Ensuite, le développement économique qui n'est possible que dans un environnement sain. Lors de sa déclaration à Luanda. Le président de la République a souligné l'importance de la diversification de l'état de l'économie angolaise et de la souveraineté alimentaire. La France encourage le renforcement des partenariats en mettant l'accent sur la formation professionnelle, le développement de filières agricoles et agroalimentaires ainsi que sur la modernisation des infrastructures dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports, notamment dans le cadre du programme chose Africa de ce que nous devons maintenant observer ce sont des résultats concrets, tels que la création d'usines et de ferme. Enfin les enjeux sécuritaires qui sont encore au coeur des préoccupations. Ainsi en est-il de la piraterie qui sévit depuis 2005 autour de la Corne de l'Afrique. Malgré une mobilisation internationale sans précédent ce fléau demeure une menace pour les transports maritimes. Rappelons que, selon la Banque mondiale les rançons ont rapporté entre 339 et 413 millions de dollars aux pirates et à leur commanditaire entre 2015. 2005 et 2012. Toutefois en 2021 et 2022 le nombre d'actes de piraterie et de brigandage maritime a diminué de façon significative au niveau mondial, avec une baisse de 15% par rapport à 2020, selon la ICA Center, basé à Brest face à la persistance du phénomène. Quelle stratégie adopter la présence des bâtiments militaires de l'OTAN a permis une diminution notable des actes de piraterie mais les eaux africaines présente encore beaucoup de dangers. Maintenant passons à l'influence grandissante de la Russie et de la Chine en Afrique, nous devons faire face à ce fait la présence et l'influence de la France en Afrique ne sont plus ce qu'elles étaient depuis une quinzaine d'années, nous avons été témoins depuis mai 2022. Des slogans antifrançais. Scandé devant notre ambassade à Pretoria où il les drapeaux bleu-blanc-rouge. Ont été brûlés. C'est le reflet d'un sentiment anti-occidental croissant en Afrique et nous y répondrons en effet face à ce changement. La diplomatie française opère un changement de posture et se réarme ce qui se traduit par plus de communication des partenaires renouveler des actions accrue vers la jeunesse et des Liens solides avec la diaspora française à l'étranger.

confond se concentre sur la côte est de l'Afrique tandis que la Russie, avec une présence plus marquée en Afrique francophone et au salles pour ça elle profite de la fin de l'opération comme cela est clairement réaffirmée par l'article 4 de la loi de programmation militaire. La réduction de la présence militaire française ne signifie ni retrait ni désengagement mais plutôt une adaptation aux évolutions des menaces et aux besoins des pays partenaires, chaque pays africains doit renforcer sa propre autonomie sécuritaire aucune ancienne base Barkhane ne sera fermé mais toutes seront destinés à former plus de militaires des pays concernés. Comme vous l'avez déclaré Monsieur le Ministre, ce n'est pas du tout un recul de la France dans ces pays. C'est une matière. Une manière d'être présent différemment. Il s'agit d'États souverain et notre présence correspond à ce. Les bases évoquée par le président correspond et ce sont celles mises en place par les accords de défense entre 2 États souverains. Il a été demandé au ministère de conduire une réflexion sur le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Gabon. Par ailleurs, le Bénin, qui semble devenir le nouveau ni du djihadisme pourrait être en train de suivre le chemin du Mali et du Burkina Faso qui se sont tournés vers la Russie suite aux manifestations contre la force Barkhane Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, comment pourrait-on imaginer la réponse constructive de la France pour préserver ses liens historiques, tout en respectant la souveraineté et les aspirations de ces nations africaines. Je vous remets. La parole est au président Pierre Laurent pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Avez la parole. Monsieur le Président Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La déclaration du gouvernement sur la politique de la France en Afrique, dont nous débattons ce soir s'inscrit dans la droite ligne du discours de chef du chef de l'État du 27 février dernier. Dans ce discours, le chef de l'État a proclamé que la France doit refuser d'entrer dans une logique de compétition qu'il faut tourner la page de l'économie de rente qu'il convient d'entrer dans une logique partenariale d'investissement solidaire. Mais le problème c'est que tous les fondamentaux dépassé de nos rapports économiques qui savent depuis tant d'années, le développement des pays africains et qui sapent aujourd'hui la confiance. Dans notre relation à l'Afrique sont aujourd'hui maintenu au mépris de tous les nouveaux enjeux du XXIe siècle. Alors que les pays africains cherche par exemple le financement de leur développement. Nous continuons de faire l'éloge de la pseudo réforme unilatérale du franc CFA qui laisse en l'état les instruments de la domination monétaire en vigueur et n'a constitué en vérité qu'une OPA hostile visant à tuer dans l'oeuf le projet de monnaie. Ouest-africaine de la CEDEAO. L'Afrique elle-pourtant on continue de parler de retrouver de la souveraineté monétaire. Mais quand j'ai interrogé dans la foulée de ce débat le gouvernement sur le stock d'or de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui est toujours détenu à 80% à la Banque de France ou la publication d'une annexe mentionné à la convention de garantie entre la Banque centrale de l'Europe de l'Afrique de l'ouest et la République française, on m'a répondu, circulez il n'y a rien à voir. Nous parlons d'être un partenaire d'avenir du développement en Afrique. Mais nous ne portons pas le faire contre l'organisation du commerce international. La nature des échanges franco-africains qui l'entrave. Les traités de libre-échange foncièrement inégaux le démantèlement des services publics et des embryons d'États social dans ces pays, la course au moins disant fiscal. Le nivellement par le bas de la protection des travailleurs, les politiques de prédation et et de Maxi bénéfices des multinationales qui agit sur place en toute impunité. Dans le cas de la France par exemple si le commerce extérieur en Afrique subsaharienne ne représentent qu'environ 2% de notre commerce extérieur. Les parts de marché, nous le savons tous sont concentrés dans les mains de quelques grands groupes qui font des affaires avec un taux de profits indécents en complicité avec des élites extraverti et corrompu au détriment de la très grande majorité des Africains. J'ai souvent dénoncé des exemples caricaturaux comme la surfacturation par des groupes français du train urbain d'Abidjan où les profits accumulés par le groupe Bolloré dans les ports ouest africains dont il est parti sans égard pour les pays concernés. Le coût pour les peuples africains du maintien de ces rapports économiques est exorbitant. Il se nomme grande pauvreté sous-alimentation maladie endémique insécurité corruption des élites migration forcée. Quand allons-nous et c'est tout cela dont la jeunesse africaine ne vole plus quand allons-nous comprendre que le rejet de la politique française, trouve ici ses ses racines profondes et ne peut être réduit au succès d'influenceurs, russes, turcs, chinois. Ou d'autres encore qu'en tireront-nous vraiment les leçons des dizaines d'interventions militaires françaises en Afrique, dont la dernière Barkhane est en vérité un échec politique lourde de conséquences. Notre politique reste à 1000 lieues des exigences populaires dans les pays africains en faveur d'une vraie souveraineté d'une 2ème indépendance comme ils disent. Exigence qu'ils expriment concrètement de plus en plus souvent. Vous ne comblerait pas ce fossé en lançant un média de propagande pour voter vanter les mérites de la politique française. N'en déplaise à ceux qui, au gouvernement et parmi nos collègues évoquent abondamment la lutte d'influence pour tout expliquer. La seule manière de combattre efficacement les fake news et les propagandes hostiles et la mise en cohérence entre les paroles et les actes de la politique française en Afrique. Si nous écoutions vraiment les jeunesses africaines. Si la France changer réellement de politique pour respecter la soif de liberté de souveraineté de développement choisi. Alors nous aurions tous à y gagner ici et là-bas car l'agenda des objectifs d'un développement durable, maîtrisé par les Africains eux-mêmes et la clé d'un véritable avenir de paix et de justice sur laquelle refonder nos relations. D'abord l'Afrique a besoin de financement massif et de création monétaire. La France doit cesser sa mise sous dépendance de la zone du franc CFA mais plus elle doit agir au plan international pour changer radicalement les règles d'attribution des DTS du FMI. Au-delà d'une réside distribution des DTS non utilisés par les pays riches qui se fait actuellement au compte-gouttes et c'est nouveau, une réforme des conditions d'démission. Des DTS devrait favoriser les critères de lutte contre la pauvreté et le financement à grande échelle de la transition économique et écologique du continent africain. Nous pourrions ainsi aider ces pays réellement comme nous l'avons à plusieurs reprises. Soyons attentifs, je constate que les Brice Brics ne reste pas inerte pour répondre à ce besoin et si nous continuons comme nous le faisons nous passerons une fois de plus à côté des besoins d'aujourd'hui dans le domaine fiscal, nous constatons que si les recettes fiscales représentent en moyenne 34% du PIB dans les pays de l'OCDE. Elles sont 2 fois moins importante dans les pays en développement, notamment en Afrique, ce n'est pas due au hasard. Les pays africains ont besoin de nouvelles recettes fiscales, et nous devrions y consacrer des efforts en cohérence avec la réalisation des objectifs contenus dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que nous avons ratifié. Et c'est au nom des propositions de ce pacte que nous renouvelons notre proposition de flécher au moins 10% de l'APD. Vers le soutien au renforcement des systèmes fiscaux de ces pays pour les leur donner des moyens budgétaires de développement et de financement en 2 gènes. Oui nous devons j'entends souvent dire. Ici, l'Afrique et notre avenir. Mais elle est d'abord l'avenir des Africains et c'est par là que tout doit commencer et qu'avec eux partenaire enfin respecter nous devrons surmonter les défis communs en matière sociale climatiques et environnementales. La France pourrait ainsi passer. D'un peu d'une politique de conquête abrupte. Et inopérante de parts de marché à trop court terme. Une politique de VRP de vente d'armes et de systèmes de sécurité. Une politique de stigmatisation hypocrite d'émigration, alors que ce sont les politiques que nous développons qui les provoque à une autre logique de rapport mutuellement avantageux de coopération repenser. En appui des choix endogène de développement de ces pays. Nous devrions encourager une industrialisation indispensables pour ces pays nous devrions Ray encourager une agro-écologie vivrières qui a largement faire ses preuves, y compris au Sahel. Plus d'eau que de soumettre les pays africains des accords commerciaux qui déstructure leur filière agricole et de pêche. Enfin si nous comprenons l'impasse de nos aventures militaires à répétition. Nous devrions. Prendre un tournant concernant les bases militaires permanentes en allant le plus rapidement possible vers leur suppression. Soyons lucides et honnêtes l'exercice par la France de ce pan important de la souveraineté des pays africains a produit globalement des résultats très médiocres dire cela n'est pas renoncer à toute coopération militaire avec les pays précités. Mais c'est accepter le refus des pays africains d'être dans une relation exclusive et dépendante en matière militaire, comme dans tous les autres domaines il faut accepter qu'ils aient une pluralité de partenaire stratégique. À défaut, nous précipiteront une évolution que nous dénoncerons peut-être avec véhémence. Oui Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, c'est dans tous les domaines, qu'il faut changer de logiciel en Afrique. J'y suis allé un peu à la serpe, je le reconnais, il faudra construire en même temps avec la Mais il faudra résolument aller vers ce changement de logiciel. C'est ce que nous ne cessons de proposer et ce que, ce que ne cesseront désormais de nous rappeler les peuples africains. Merci, La parole est à notre collègue Joël Guerriau pour le groupe les indépendants République et Thierry. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires étrangères et de la défense. Mes chers collègues. Le 15 juillet 1959. Le général de Gaulle ouvrait ici même la première session du Sénat de la communauté.

À peine un an plus tard au printemps 1960 la fin prématurée de la communauté nous renvoie au discours du général De Gaulle et je cite. La grande chance de la paix et de la civilisation, c'est que les hommes, les enfants de l'humanité qui dispose des moyens voulus. Apportent leur aide à cette humanité tout entière. 60 ans plus tard, nous souhaitons entretenir lien d'estime et d'attachement réciproque avec le continent africain. Vous l'avez rappelé Madame la Ministre nous tentons au mieux de nos capacités de contribuer à apporter notre aide. Lorsqu'elle est souhaitée pour résoudre les crises de ces pays que ces pays rencontrent. Plus de la moitié de l'aide publique au développement de la France est consacré au continent africain. La coopération décentralisée des collectivités françaises participent à construire des infrastructures des puis des routes, des écoles des dispensaires afin d'améliorer le. Des populations et ce faisant, nous compris. Bon à réduire la pauvreté et ses conséquences conflictuel notre engagement bien sûr ne s'arrête pas là. Vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre, nous participons depuis de nombreuses années à des missions de maintien de la paix. La France a notamment répondu présentes en 2013 lorsqu'elle a été appelée pour empêcher des djihadistes de prendre Bamako 53 soldats français ont pire au Sahara au Sahel lors de ces opérations et je veux bien sûr leur rendre hommage ce soir avec une pensée pour la famille et pour leurs camarades. Malgré la force c'est la constance de notre engagement, notre pays fait l'objet depuis environ une décennie de campagne. Propagande destinée à attiser la haine à notre égard. La Russie comptant parmi les meilleurs spécialistes de la désinformation. Nous n'avons pas été surpris de voir la milice Wagner intervenir en Centrafrique, puis au Mali. La France encore davantage depuis le Brexit. Assume un rôle moteur dans les opérations de maintien de la paix lancée par l'Union européenne. Nous ne pouvons cependant pas être les seuls à supporter cette charge. Assez modérément soutenue tant par les gouvernements locaux que par nos partenaires européens. Notre pays a progressivement réduit son engagement en Afrique. Force est cependant de. Que la prolifération de mouvement islamiste l'intervention de la milice russe et le piège de la dette chinoise ouvre de sérieux motifs d'inquiétude. Avec la croissance démocratique démographique et le dérèglement climatique. En toile de fond l'Afrique est exposée au risque de grave Christ. Nous assistons aujourd'hui à une véritable crise des institutions dans certains États africains. Les récents événements au Soudan confirme cette triste perspective. Tout comme la famine qui menace la Corne de l'Afrique. Plutôt que de préparer l'avenir. Beaucoup ont malheureusement été détourné de la réalité par une idée qui continue de faire couler beaucoup d'encre. La Françafrique bouc émissaire de tous les maux. Ce comportement trouble une appréciation correcte. Que des faits politiques couvrant par des mensonges l'incapacité de dirigeants à répondre aux attentes de leurs peuples. Le pouvoir se concentrant les mains entre les mains d'un président au lieu de junte qui use et abuse de son pouvoir. Les faits sont cependant bien éloignées des thèses imaginée par des agitateurs sur. Sur les 2 rives de la Méditerranée. La raison en est simple, l'ensemble du continent africain représente environ 5% du commerce extérieur français en 2022 et ce chiffre fait voler en éclats le fantasme de l'eldorado. Le 1er partenaire commercial de l'Afrique et désormais la Chine le poids de la France ne cessent de s'amenuiser à mesure que d'autres puissances prennent leur essor. C'est une réalité à laquelle nous devons nous adapter cette réalité autre aussi composer de nouvelles amitiés tout comme l'Afrique du Sud, l'Algérie qui ne cache. Plus sa proximité avec Moscou à la mené des exercices militaires avec l'armée de Poutine et refuse dans le même temps de délivrer des laissez-passer consulaires nécessaires au retour de. Les Algériens expulsés par la France, elle n'est pas la seule à s'être égaré après plusieurs couches. Putsch le Mali s'enfonce dans la crise préférant répondre par la force aux carences de son état. Ce ne sont là que quelques exemples, ils sont autant de signes d'une tendance qui voit l'influence occidentale reculer sur le continent africain. Nous n'avons-nous pas les mêmes valeurs que la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping, les gouvernements africains. Sont libres de nouer de nouveaux partenariats libre et donc responsable il leur reviendra d'assumer l'ensemble des conséquences qui en découleront. Dans cette nouvelle configuration, il est nécessaire d'ajuster la politique étrangère de la France, faut-il continuer nos efforts en poursuivant les mêmes orientations avec la même intensité. En avons-nous encore les moyens. Éprouvés par la crise de la Covid nos finances publiques sont dans un état préoccupant. Elles sont d'ores et déjà mobilisés par le retour de la guerre en Europe. L'invasion russe de l'Ukraine a fait prendre conscience aux Européens de la nécessité de prendre en main leur propre sécurité. Les efforts budgétaires consentis par les gouvernements du continent sont conséquents et vise à préparer nos armées a désengagement de haute intensité avec des moyens limités, la concertation avec nos partenaires européens est encore plus nécessaire. La France sait depuis longtemps qu'il est dans l'intérêt de l'Union européenne de se préoccuper du devenir du camping africain certains États doivent encore être convaincu. La population qui compte aujourd'hui plus de 1 milliard d'individus pourrait passer à 2,4 milliards d'ici à 2050 dans le même temps l'accroissement de population peut intensifier la gravité des crises, celle qui ne trouvent pas de solution locale génère des déplacements de population qui elle concerne directement notre continent européen. Le groupe les indépendants. C'est-à-dire que les ambitions de la politique étrangère de la France en Afrique doivent être proportionnées aux des moyens dont nous disposons à cet effet, nous saluons la décision du président. Relatives à la cogérance de bases militaires avec les pays dont nous partageons les objectifs. Il conviendra également de repenser notre relation avec l'Afrique sur les plans sécuritaire migratoire économique également de retrouver des instances de dialogue et d'échange. À l'instar de l'Union pour la Méditerranée. Il nous paraît. Ensuite nécessaire de concentrer nos efforts sur les pays qui partagent nos valeurs et se montre solidaire. Rappelons que 7 pays dont l'Érythrée et le Mali. À l'ONU, ont refusé de condamner l'agression. Son russes en Ukraine. Nous n'avons pas que des amis parmi les dirigeants africains dans la nouvelle configuration et il nous semble qu'il est important d'investir en faveur de nos alliés, en veillant à ne pas renforcer nos adversaires. Cela implique une stricte sélection des pays et des projets auxquels nous consacrons notre raide. Qu'il s'agisse de la vie de nos soldats ou 2 milliards d'aides publiques également libre et indépendante. La France doit agir au mieux de ses intérêts pour cela une approche paraît adapté avec 2 axes essentiels à nos yeux la réciprocité avec une entente cordiale. Merci. La parole de notre collègue André guignol. Pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Monsieur le Président Madame la Ministre. Monsieur le Ministre. C'est le président de la commission mais chaque collègue. L'Afrique est le continent ne tous les défis climatiques. Démographiques et économiques. Il est aussi celui de tous les âges, pour ne pas dire de toutes les convoitises. L'intérêt de la Chine et de la Russie ont permis de sortir l'Afrique de son face à face avec l'Europe mais à quel prix. S'agissant de la Chine. La masse d'argent qu'elle a déversé sur de nombreux pays africains a crée une relation asymétrique qui n'a pas forcément apporter le développement attendu bien que Pékin avec Pékin prétendent depuis 2 ans, ouvrir une nouvelle ère pour lui aux relations financières plus soutenable avec ses partenaires. Quant à la Russie, on le sait, elle y mène également sa stratégie d'influence avec des moyens peu conventionnels. Si l'on songe au travail de sape mené par le groupe privé Wagner sur le thème de l'Occident décadent et toujours à de domination. qu'il en soit, les moyens, quelles que soient les moyens. Cette stratégie est payante pour Moscou et on a vu l'abstention, de plusieurs pays africains sur les résolutions condamnant l'agression russe en Ukraine. L'abstention du Gabon entre autre sur ce dernier texte porté par Paris est assez éclairante. Face à cela, que peut l'Europe. Que peut la France qui traîne dire derrière elle le poids de l'histoire coloniale des difficile. Le mouvement de deal de Libération et de la politique du pré-carré qu'elle a installé dans les années 60. On en connaît les conséquences dans certains pays, les relations avec la France demeure hélas passionné ou traumatiques. Pourtant depuis bien longtemps. Sans renier le mémoire aux communes et les réparations qui en découlent. Nos présidents successifs ont appelé à regarder l'avenir plutôt que le passé. De son discours de à l'université de Ouagadougou jusqu'à ses récentes déclarations dans le cadre de sa dernière tournée diplomatique d'un 4 pays africains le président Marc. Emmanuel Macron n'a cessé de soulever la fin de la Françafrique et la nécessité de refonder une relation équilibrée. Comment ne pas partager cette volonté. Par la force des événements, il ne resterait heureusement plus grand chose de la Françafrique. La fin du franc CFA. En quelque sorte le témoignage symbolique. Aujourd'hui, mes chers collègues. Quelle page ouvrir avec l'Afrique pour construire une nouvelle ère dans le contexte géopolitique que j'ai évoquées au début de mon propos, ainsi que au regard des grands défis que nous ne pouvons affronter qu'ensemble. Il me semble que la première règle consisterait à toujours demander à nos partenaires ce qu'ils attendent de nous. Il faut bien sûr pour cela que la relation soit franche et sincère. Je le conçois. Et ce n'est pas aisée, mais le président Macky Sall ne sait pas. C'est ce type pas servi du sentiment antifrançais pour mieux justifier son maintien. À la tête du Sénégal. L'instabilité politique aussi peut être prendre de bonnes intentions compliqué. Nous l'avons vécu au Mali, la France directement appelé en 2013 par Bamako pour stopper l'avancée des troupes armées islamistes a été prise a été prié de partir de 20 ans plus tard par la junte installé au pouvoir. De notre côté, sur le plan diplomatique il faut clairement éviter tout geste qui pourrait apparaître comme un adoubement de tels ou tels dirigeants putain certains États sont encore politiquement très fragile et versatile. Sur le plan sociétal. Je crois aussi qu'il ne faut pas surestimer le rayonnement de la France. Même si le français langue de culture pour reprendre les propos de Léo pour Senghor est encore bien vivace grâce aux instruments de la francophonie. Cependant restons humbles et sur ces l'échange mutuel dépoussiéré des vieux démons. Essayons d'orienter toutes nos politiques de coopération sous l'Arc de la coproduction. C'est sans doute ce qu'attendent les nouvelles générations. Qui veut le prendre en main leur propre développement et qui ont à notre égard des aspirations égalitaires plus prégnante. Cela est vrai. Même sur le plan militaire. Nos accords de coopération, de me mettre davantage l'accent sur les aides à la formation et sur les équipements des armées locales. L'envoi de troupes doit être le dernier recours ou se fondre dans une alliance équilibrée. Cela ne doit pas empêcher pour autant le maintien de nos bases militaires essentiel et pour notre stratégie de défense ainsi que des échanges de renseignements avec nos partenaires africains. Nous allons un partage. Nous avons en partage les enjeux sécuritaires dans la lutte contre l'infatigable terrorisme islamiste. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, je crois que c'est bien le sens de la volonté du chef de l'État qui a souhaité lors de sa dernière allô. Christian le 14 juillet une offre militaire française rénové en Afrique. Mon groupe au partage, en tout cas le principe d'une présence partenariat le plus discrète et de, de préférence dans le cadre de multilatéral autant que possible. Ça, je dis, s'agissant de la coopération économique, là encore il faut se demander quels sont aujourd'hui les besoins de nos partenaires. L'Afrique ne doit pas être seulement le pourvoyeurs de matières premières comme l'a très récemment rappelé Azali Assoumani, le président en exercice de l'Union africaine. La Banque africaine de développement, avait publié l'année dernière, l'année dernière, l'indice d'industrialisation de l'Afrique 2022, indiquant que les économies les plus industrialisés d'Afrique était celle qui avait produit le plus d'efforts pour s'éloigner de la dépendance vis-à-vis des industries extractives. Et pour se Et pour se tourner vers des secteurs à valeur ajoutée. Dans ces conditions les entreprises françaises et en particulier les PME ont tout intérêt à prendre ce virage et investir dans ce sens. Les pays anglophones, avec lequel nous n'avons pas d'antécédent, si je puis dire. Doivent aussi retenir un peu plus fort. Attention sur les investisseurs français. Enfin, mes chers collègues parce que l'Afrique est aux portes de l'Europe, nous devons aussi maintenir un lien fort avec plusieurs de ces pays pour la gestion du flux migratoire. L'explosion démographique du continent, nous invite à regarder cette question avec ouverture car c'est qu'a rien n'arrêtera ce mouvement. À cet égard au-delà de nos accords bilatéraux sur le problème migratoire, il revient à l'Union européenne de travailler au plus proche. Je veux dire, oui les institutions régionales africaines pour un peu plus effective de l'approche globale, adoptée en 2005 par l'Union européenne basée sur 3 axes. La promotion, la promotion de la mobilité et la migration légale la prévention et la lutte contre l'immigration clandestine et l'optimisation du lien entre migration et développement. Garderont aussi à l'esprit que l'Afrique ne ne doit pas être privée de ses talents indispensable à son développement. L'immigration choisie a ses limites. Il est temps de penser notre coopération interne gagnant gagnant. Alors, mes chers collègues. Il est évident que la France doit écrire un nouveau récit avec le continent africain et faire la démonstration de son utilité car notre pays a une expertise et une valeur nécessaire à la défense des intérêts de l'Afrique, dont certains sont aussi des. Autre je vous remercie. Merci. La parole est maintenant au président Guillaume Gontard. Pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le 9 novembre 2022, le président de la République a annoncé la fin de l'opération Barkhane. Près de 10 ans après le déploiement de l'armée française au Mali. 10 ans de présence au Sahel et un seul vote du Parlement en 2013. Depuis, malgré les évolutions militaire considérable qu'ont connu les différentes opérations au Sahel. Pas une seule fois le Parlement n'a pu exprimer son avis. Toutefois, les décisions ont été prises de manière unilatérale au sommet de l'État même si vous nous avez fait la grâce d'un débat sur la possibilité d'un retrait français du Mali. En février 2022. Et que vous nous fait la grâce de celui-ci. La politique africaine de la France demeure une chasse gardée du pouvoir exécutif. Cela n'est pas gage d'efficacité, puisqu'il est délicat de trouver une quelconque satisfaction au bilan de la décennie écoulée. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore forcé de constater que jamais la position de la France en Afrique n'a pas réussi précaire. En préambule, quel bilan pouvons-nous tirer de l'opération Barkhane. Je voudrais tout d'abord au nom du groupe écologiste renouveler mes pensées pour les 59 militaires morts au Sahel depuis 2013. Leurs familles et leurs proches. La reconnaissance de la nation est éternel. Nos forces armées se sont déployées au Mali en 2013 avec pour objectif d'empêcher une progression de la menace djihadiste. Si pour Emmanuel Macron. L'opération Barkhane n'est pas un échec, nous pouvons tous ici convenir du fait que la menace djihadiste est loin d'être éradiquée. Alors que les jihadistes avaient reculé en 2014, ils sont aujourd'hui bien présent dans le nord et le centre du Mali, mais aussi au Burkina Faso, au Niger ou encore en Côte d'Ivoire. Et situations politiques des pays concernés par l'opération Barkhane sont préoccupantes. Après plusieurs coups d'État récent le Mali et le Burkina Faso, sont aujourd'hui sous l'emprise de junte militaire. Nous le craignons sans solution politique pérenne les opérations militaires ont peu de chances d'aboutir à une situation stable depuis notre retrait du Mali en 2022 et du burlesque, du Burkina Faso, pardon en 2023. Les djihadistes s'engouffre dans le vide laissé par nos forces armées. L'opération Barkhane montre clairement les limites d'une intervention extérieure purement militaire, sans aucune vision de sortie de crise. La situation chaotique de ces pays et de bien d'autres en Afrique couplée avec un sentiment anti-français de plus en plus prégnant ouvre la voie à l'influence russe et en particulier à la milice Wagner aujourd'hui présente dans 17 pays africains. La relation étroite de la France avec le continent africain s'est abîmé le sentiment anti-français a progressé à grande vitesse ces dernières décennies. Mais pourquoi. croissante croissante pardon de puissances étrangères, cherchant à instrumentaliser le rejet de la France, l'explique, mais seulement en partie. C'est notamment le manque important de transparence des opérations militaires françaises qui est mis en cause. Comment les peuples et gouvernements africains peuvent-ils nous faire confiance. Quand nous prenons des décisions sur l'avenir de leur pays sans leur consentement. Ce modèle d'intervention militaire paternaliste qui ça. Ce qui n'associe pas ou peu la décision des gouvernements des pays théâtres d'opérations a fait montre de toutes ses limites. Une nouvelle fois. Il paraît impensable à l'avenir d'envoyer nos troupes dans des pays sans débouché politique tangible ou sans association étroite sur la durée avec le pouvoir politique en place. Nous devons absolument être plus transparents sur nos actions et reconnaître nos bavures et horreur comme le dramatique bombardement d'un mariage le 3 janvier 2021 au Mali. Les peuples africains reprochent également à la France une indignation à géométrie variable concernant leurs dirigeants selon leur degré de coopération avec Paris. Et a raison pourquoi dénoncez à juste titre la dictature militaire au Mali mais soutenir Idriss débris débit par contre président du Tchad pendant 30 ans, puis son fils, placé au pouvoir après sa mort, le respect de la volonté des peuples et des droits humains doivent être notre boussole. Alors que les effectifs de l'armée française sont réorientés au Niger et au Tchad là où demeure certains intérêts stratégiques vitaux comme la fourniture d'uranium de nos centrales nucléaires. Il est plus que clair que nous devons bâtir un nouveau type de coopération avec le continent africain. Les accords de défense comme les partenariats économiques doivent être conclue dans l'intérêt des peuples tout en prenant garde à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des pays. En parallèle, il nous faut continuer à soutenir le développement du du continent et renforcer notre solidarité avec les pays les plus pauvres notamment via notre aide publique au développement. Si des efforts notables ont été effectués depuis le vote de la loi de programmation, il y a 2 ans. Nous rappelons avec force la nécessité de contribuer au développement par des dons Directs et non des prix ces derniers conduisent à prioriser les pays à revenu intermédiaire plutôt que les pays pauvres. L'aide apportée par notre pays doit être beaucoup plus ciblées et. Garantir la sécurité la subsistance à travers des réseaux locaux est une autre manière de lutter contre les terroristes qui bien souvent assoit son influence en soupe venant aux besoins des populations. Nous devons ce juste retour qu'à notre dette envers le continent africain est immense mais nous devons aussi accompagner l'Afrique dans un développement qui se doit immédiatement d'être durable. Il faut davantage conditionner les aides versées au respect des droits humains démocratiques, sociaux et écologiques notamment les droits des femmes et ceux des peuples autochtones ne me demandons enfin que l'aide si opportune. Opportunément accordé aux réfugiés ukrainiens sur notre sol intègre nos comptes sociaux et ne soient plus comptabilisés comme un effort d'aide publique au développement. En plus de l'APD, il est nécessaire d'annuler les dettes de certains pays africains, notamment les dettes contractées par des dictatures dans le seul but d'enrichir le clan au pouvoir ou d'engager des actions qui vont à l'encontre de l'intérêt général. Tout cela est indispensable pour anticiper les futures décennies nous savons les pays les plus au sud, les pays les plus pauvres vont subir et subissent déjà les conséquences les plus graves du réchauffement climatique. Sommes-nous prêts à accueillir les futurs réfugiés climatiques qui arriveront par millions en Europe. Nous peinons déjà à accueillir dignement les réfugiés qui entrent sur notre sol, durcir les politiques migratoires déjà en vigueur ne sera d'aucun secours face à de tels mouvements de population. Allons-nous continuer à laisser des entreprises françaises mener des projets climaticides comme le nouvel oléoduc de Total en Ouganda ou en Tanzanie qui émettra 379 millions de tonnes équivalent CO2 en 25 ans, soit 216 millions de liaison aérienne Paris-New Paris-New York, les scientifiques sont pourtant clairs, si l'on veut atteindre zéro émission nette en 2050, plus aucun projet fossile n'est possible. En plus du risque climatique avéré. Les ONG dénoncent déjà plusieurs cas de violations des droits humains de Total, en Ouganda et en Tanzanie. Cela me fait dire que qu'il est plus que temps de renforcer l'application de la loi sur le devoir de vigilance des entreprises de 2017 voire 2 musclé en transformant le devoir de vigilance en obligation de vigilance avec une responsabilité accrue des entreprises et des opérateurs publics intervenant à l'étranger. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes tous d'accord sur le constat, la politique africaine de la France est à un tournant. L'occasion d'adopter une toute autre attitude vis-à-vis des peuples africains et de faire primer le respect mutuel, la coopération pour accompagner le développement social et écologique du continent africain. Merci. La parole est maintenant. Le collègue Stéphane Ravier pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

dans la politique étrangère de la France en Afrique pour la déclaration de ce jour où le confirmer l'importance de cette question par l'exécutif. Mais malgré cet investissement de votre temps de notre argent et de nos coopérants civils et militaires depuis plusieurs années la défiance s'accentue la francophobie progresse et nous perdons en influence sur tout le continent, continent, pourtant le plus francophone de tous de ceux-là vous en être en partie responsable en relayant le postulat culpabilisateur qui qui repose sur le mythe du pillage colonial vous saborder les efforts concertés de notre politique d'influence, ce n'est pas le cas des autres puissances coloniales qui ne pratiquent pas cette auto-flagellation. J'en veux pour preuve nos anciennes colonies, toujours francophones et du Togo et du Gabon. Ils ont rejoint le comment sont 2022 la France doit cesser de se désigner elles-mêmes comme un bouc émissaire ce masochisme injustifiée ne saurait servir de base à une relation fructueuse entre la France et les pays africains, la 2ème erreur et celle de vouloir exporter la démocratie comme une recette universellement transposable. Nous avons vu ce que cela avait donné par le passé en Libye et ailleurs chaos aggravé chez eux importé chez nous la 3ème erreur c'est celle de refuser de faire de la politique, en vous cantonnant à des partenariats avec le monde de la culture de la jeunesse. La société civile comme seul horizon par idéalisme vous renoncez à faire de la France une grande puissance de plus vous faites croire que notre recul militaire est un choix, alors qu'il est majoritairement contraint par les États africains qui nous mettent dehors la 4ème erreur c'est celle de refuser d'adjoindre à l'aide publique au développement. Une injonction de puissance et une et une exigence de réciprocité, sans lesquelles nous subissons la double peine financière et migratoire La 5e erreur c'est celle de la suppression du corps diplomatique, elle sonne à la fin d'une tradition africaine au sein du Quai d'Orsay, la perte d'un réseau d'un savoir-faire et des connaissances acquises durant de nombreuses décennies. On a vu les conséquences et des négociations improvisées par le politique. Nous sommes en froid avec tous les pays du Maghreb viré du Sahel et fâchée avec l'Afrique centrale. Dans le même temps, toutes les grandes puissances et s'implante massivement et durablement en Afrique. La Chine, l'Iran, la Russie, la Turquie, les pays du Golfe au Gabon 70% de la 2ème plus grande forêt du monde après l'Amazonie appartient aux chinois pendant que Wagner s'occupe du militaire. Pékin s'affairent à la coopération économique, enfin avec le départ de la force Barkhane. Nous avons perdu la main dans la lutte en amont contre l'immigration illégale et les terrorisme islamiste. Aujourd'hui, le président tunisien parle de grand remplacement avec l'Algérie et le Maroc ils contrôlent désormais le robinet d'une déferlante d'une déferlante migratoire qui enfle chaque année un peu plus au vu de l'explosion démographique du candidat continent africain il y a une impérieuse nécessité de stabilité politique et de développement économique en Afrique et de fermeté en Europe, la lutte contre et trafic d'être s'humains devient un marché juteux. Au même titre que les trafics de drogue et qui s'intensifie du sud vers le nord et en conclusion pour faire écho aux propos pertinents exprimée par le président Cambon. Je vous rappelle Madame le Ministre et Monsieur le Ministre, que pas que parier sur l'Afrique commence par parier sur la puissance de la France. merci. La parole est. Maintenant après la somme des orateurs des groupes. Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et ensuite au ministre désormais comme vous souhaitez. Merci Merci monsieur prudent. Mesdames. Et messieurs les sénateurs. Merci à chacun d'entre vous 2 de vos interventions et je crois que la première chose que je souhaiterais dire c'est que nous faisons souvent un constat partagé sur les enjeux sur les défis que représente le continent africain. Les pays africains dans dans leurs relations avec nous dans la révolution et je crois. Constat partagé également. Du fait que nous devons continuer à évoluer transformer. Notre approche. Monsieur le Président Cambon quelques remarques. Partielle. Dans vos points ont été nombreux. Mais je voudrais revenir très très brièvement sur les relations commerciales que vous avez évoquée et dont j'avais tenu à dire par précaution que oui l'Afrique s'était diversifié comme nous même nous faire scission de partenariat. Mais que nos exportations notre présence présence économique est plus forte qu'auparavant, ils ont progressé donc en en volume et en parts de marché, ça n'est pas la même chose. Chacun peut retenir. Ce qui lui semblera le plus pertinent, je nous fais donc aucun reproche président. Je reviendrai plus longuement sur. L'expression souvent entendue et que je crois trompeuse en grande partie de sentiment anti-français. Je souhaiterais qu'on fasse attention à cette expression parce que elle induit des choses qui ne sont pas et monsieur le sénateur, vous l'avez souligné, il faut distinguer, me semble-t-il le discours antifrançais. Du sentiment antifrançais et ce que nous voyons souvent c'est un discours anti-français qui se. Répand qui se répand. Pas tout seul mais je l'ai déjà dit et qui a joué. Oui un rôle majeur dans dans le basculement du Mali dans le basculement. Peut être du Burkina Faso. Mais il ne faut pas confondre l'un et l'autre c'est le recours à Wagner, par les autorités. De fait, de la RCA ou. Au Mali, issu de coup d'État qui entraîne la diffusion d'un discours antifrançais et en d'autres termes. Ça n'est pas le le sentiment anti-français qui ferait partir à la France c'est. Plutôt l'arrivée de Wagner conviée par des putschistes, comme le disait le ministre des armées. Qui fait venir la prédation des exactions et le discours anti-antifrançais. Nous avons décidé de réagir. Ne nous réarmer les moyens sont en augmentation et aussi de dénoncer. Ces manipulations de l'information. Monsieur le président vous avez aussi dit je crois vous soutenir parfaitement que nous devons assumer nos intérêts les assumer de façon. Honnête, respectueuse décomplexé d'égal à à égal comme partout dans le monde et je partage le constat que vous faites sur l'influence. Nous augmentons. Pour faire face à ces nouveaux enjeux nos crédits nos demande au crédit de communication et nos crédits dans les. Services culturels. Disons qu'on appelle maintenant influence mais les CKAC dans notre jargon. Nous allons également augmenter, vous avez vu des annonces faites par le président de la République après la réunion du comité. Du Conseil pardon présidentiel du développement. Donc nous avons décidé d'augmenter notre expertise technique de plusieurs centaines. De TI. D'ici 2027. Je reviendrai sur. Certains des aspects madame la sénatrice Carlotti que vous avez évoqué d'abord la trajectoire de l'APD oui la loi d'août 2021, vous le savez mieux que moi, fixent des niveaux mais ils fixent des niveaux jusqu'cette année. Ensuite, elle fixe des objectifs, ce n'est pas la même chose. Un objectif n'est pas impératif. D'autre part je dois à nouveau faire remarquer que notre APD a augmenté en volume. Je ne connais pas d'autres pays qui a augmenté son aide à l'Afrique en volume, je le disais et d'une façon plus générale, la France a augmenté a augmenté de 50% son aide publique au développement, entre 2017 et 2022 donc le volume de l'APD continue d'augmenter. Merci madame la sénatrice des éloges que vous rendez à un haut diplomate. j'y suis sensible, vous le savez bien mais je ne crois en rien que notre action diplomatique soit affaibli. Lorsque le président de la République décide d'augmenter les moyens du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères décide d'en augmenter les emplois cette année pour la première fois depuis 30 ans et donc après 30 ans de déclin ou décide d'en augmenter les moyens budgétaires sur une trajectoire pluri-annuel. Nous menons jusqu'à 2027 et pour le reste, madame la sénatrice, non seulement nous n'avons pas la nostalgie. Du passé où la nostalgie de relation. Exclusive mais notre relation a changé dans les fêtes nos sont des partenaires nous sommes respectueux des partenaires que nous avons sur le continent africain. Nous assumons nos intérêts je lisais et nous nous tournons davantage vers les défis communs les grands défis globaux. Le climat d'insécurité alimentaire et tant et tant d'autres choses. Monsieur le sénateur, qui a dit que vous avez. avez. Évoqué l'influence de la désinformation, je n'y reviens pas, mais c'est un point important, la politique des visas. Monsieur le sénateur est une politique menée conjointement par le ministère de l'Intérieur. Et par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ou plus exactement, dit le décret d'attribution du Ministre de l'intérieur par le ministère de l'Intérieur conjointement avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous ne nous empêche pas de piloter ensemble avec Gérald Darmanin, nous avons tenu un comité de pilotage tout récemment nous permettant de constater que la politique des visas permet de protéger nos intérêts à de nombreux égards, mais est aussi une politique qui permet l'attractivité de notre pays point que nous avons développé l'un et l'autre en confiant. À monsieur Hermelin. Le rapport dont j'espère vous pourrez bientôt prendre connaissance avec l'appui des 2 inspection générale. Nous suivrons ces recommandations et nous augmenterons également les les moyens humains dans. Nos consulats. Merci de mentionner aussi monsieur le sénateur, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le ministre des armées en parlerait mieux que moi mais cela traduit en Côte d'Ivoire, notre volonté de renforcer les capacités des partenaires. Madame la sénatrice Duranton. Qui est là. Merci madame la sénatrice. Et merci d'avoir souligné. Vous aussi vous avez parlé de virage, je crois, la rénovation de nos relations avec le continent africain. Tout le monde ne l'a pas pas fait donc je vous en suis reconnaissante. Je crois qu'il faut rappeler aussi l'intensité comme vous l'avez fait de notre travail diplomatique avec les pays africains pour relever ces défis communs, nous l'avons fait par exemple avec Le Guen Summit. Au Gabon, tout récemment, ou par exemple, nous le ferons à la fin de ce mois avec le sommet sur le nouveau pacte financier donc merci aussi de reconnaître ses efforts. C'est un processus constant. Ils doivent se poursuivre. Nous allons aussi continuer de nous réarmer comme on dit pour accroître nos capacités d'affluence. Il y a encore beaucoup à faire, nous, nous le savons mais nous y sommes déterminés. Monsieur le sénateur, Laurent. J'ai le regret et je parle sincèrement, d'être en désaccord avec vous sur un certain nombre de points. Par exemple vos affirmations sur le franc CFA qui me paraissent inexactes parce que si nous garantissons. Toujours la parité avec l'euro, à la demande des pays concernés l'obligation de centralisation des des réserves de change est terminée, elle a donc disparu. Il faut le savoir et en prendre note pour Me son logiciel si vous me le permettez au goût du jour. Désaccord aussi sur ce que vous avez dit sur nos entreprises. Le nombre de filiales. D'entreprises françaises a augmenté non pas diminué donc il n'y a pas que le grand capital. Vous n'avez pas prononcer l'expression qu'il serait présent en Afrique mais nous avons au moins un point d'accord monsieur le sénateur. Oui les pays africains sont nombreux à avoir besoin. De financement accru. Donc c'est l'un des objectifs de ce sommet des 22 et 23 juin, que de permettre un nouveau pacte financier mondial et notamment. Vous le verrez. La France, il plaidera pour une augmentation des droits de tirage spéciaux. Augmentation qu'elle a elle-même pratiqué, nous avons tenu nos engagements 2021 et mobilisé plus de 4 milliards de dollars de DTS pour les pays vulnérables. Monsieur le sénateur gueule a évoqué la Russie et aussi la Chine. Je pensais simplement je m'arrêterai là. Sur. Ce que nous voulons faire dans le cadre de ce sommet des 22 et 23 juin. Auquel la Chine sera présente est représenté par son Premier ministre, donc un niveau de participation important ce qui nous permettra de débattre aussi de la question de la dette. De points tout à fait partiel. Pourrait prendra. De sujets évoqués par le sénateur Gontard au Tchad Monsieur sénateur nous ne soutenons aucun régime nous soutenons comme tous les pays de la région une transition une transition dont nous souhaitons qu'elle mène à des élections. Et en fait en Ouganda. Je dois vous rappeler que. Si Total est en activité ou à des projets dans un certain nombre de pays africains. Il n'y a pas de financement de l'État, ni même de garanties apportées par la France aux actions de sociétés privées commerciales. Merci monsieur le président. Merci mesdames et messieurs les sénateurs. S'il m'est permis de le faire. L'organisation de ce débat parce que ce qui me frappe en un an. J'occupe ses fonctions mise c'est que malheureusement. Les questions africaines occupent désormais trop peu de place dans le, dans le débat démocratique globale. Et que ce débat même nuitamment. Et même avec une représentation proportionnée. Sur l'ensemble des des bancs nous permet quand même de le faire et de le faire pour. Le notre opinion publique de le faire pour la presse et de le faire aussi, on le sait pour les partenaires africains qui regarde. Évidemment ces débats. Mais si Monsieur sortie mal je je le dis. Je le pense vraiment sincèrement. Eh bien c'est pour c'est. Pour ça que vous êtes présent. En fait je m'en félicite. Et en tout cas c'est pour ça aussi que nous répondons bien volontiers. Hein vous différents interpellations. La ministre a tout dit, qui me. Qui m'ont marqué dans les différentes interventions qui au fait. Nadal au fait si on n'y prête un peu l'oreille semble toutes se ressembler dans le constat. Vous me direz. Nous nous aussi. Et de fait c'est pas le constat qui est le plus difficile à établir, surtout quand l'histoire est faite et quand l'histoire est terminée parle notamment pour mes affaires militaires, et pour les sujets il y a Barkhane j'ai reviendrait mais au fond quand on creuse un peu, on s'aperçoit quand même que ce sont des interventions qui sont au fond très différente dans l'approche de ce que doit être la politique française en Afrique, c'est d'ailleurs enfin démocratiquement et à la question du président Gontard sur la confiscation. D'un débat politique ou parlementaire sur ces sujets. Moi je pense, considère qu'il faut qu'il ait lieu sur le 15 jours de débats à l'Assemblée nationale sur notre programmation militaire. Je pense que c'est intéressant de voir à quel point justement un certain nombre de formations politiques sont à ce point. Non cohérentes parfois avec leur histoire, parfois avec différentes prises de position récentes récentes sur l'Europe sur le temps sur le franco-allemand sur l'aide à l'Ukraine et je pense que au contraire c'est bah si je fais 15 jours à l'Assemblée, je peux vous assurer que beaucoup de formations politiques sont très des accès entre elles y compris dans des alliances électorales. Récentes et et que donc je trouve que c'est intéressant de le faire et sur la question africaine n'y échappe pas et je pense qu'au contraire on ne sort de l'ambiguïté qu'elles sont propres détriment comme aurait dit le cardinal de Retz, c'est je pense qu'au contraire c'est sain de le faire. Ce qui m'amène à quatre remarque. La première alors Madame la Ministre Carlotti merci pour le le l'ensemble du tableau que vous avez dressé. Vous trouvez un peu dur sur Takuba.

C'est faux, ils ont répondu présent que les partenaires européens aujourd'hui, y compris des pays. Monsieur le Ministre, qui n'avaient pas l'habitude d'engager leurs forces en OPEX et qui parfois ont des parlements qui leur ont toujours refusé l'ont permis aujourd'hui en sont quand même satisfait de l'avoir fait et ont une forme de fierté que d'avoir contribué à la force C'est que le groupe socialiste ne croit plus. À l'Union européenne en la matière. Non mais j'en fais exprès je je dis juste que. J'en dis juste que. Merci Takuba de ce point de vue à fonctionner. Et si je regarde de près, mais je serai prêt à revenir en commission, le cas échéant, y compris sur des opérations militaires très précises qui ont été menées avec le timbre de Takuba sur des groupes terroristes armés. Pour le coup le c'est mal, le cas échéant lors d'une prochaine audition pourrait il revient devant vous mais enfin, il y des opérations militaires qui ont bien fonctionné. Si on va de la de de Takuba mais j'aimerais bien dans un instant, on a aussi d'autres missions européennes qui n'ont pas fait l'objet de discussions potentiel Atalante mérite quand même d'être signalé. On a parlé pratiquement pendant 3h sans parler de de, on n'a pas le temps de tout traité bien sûr mais de piraterie. De de évidemment de liberté d'accès maritime de pêche illégale. On sait que dans le Golfe de Guinée. C'est un enjeu majeur à l'approche de la Somalie, c'est pareil qu'évidemment ces sujets se se rencontrent parfois avec les sujets liés au terrorisme que dans d'autres routes de navigation commerciale. C'est malheureusement le sujet de Wagner qui peut être rencontrés donc on, on est dans une approche militaire. On est toujours dans une approche très terrestre. Je crois qu'on a on a tort de d'oublier moi le 1er d'ailleurs ce que je ne l'ai pas fait la tribune donc je je le confesse bien volontiers mais d'écarter les coopérations et les missions. Maritimes la sénatrice durant, on l'a fait depuis d'ailleurs c'est plus une mission de l'OTAN. C'est devenu une mission porté par l'Union européenne, sur laquelle la France elle est grandement contribué. On pourra y revenir, mais ça pour le coup, si on est à l'écoute des besoins des pays africains, il est clair que les besoins en matière maritime, ce sont des besoins qui sont croissants et sur lequel au fond ce sont quand même beaucoup les Européens ne des agendas de sécurité en miroir avec la mer Méditerranée ou le Detroit de Gibraltar, qui peuvent être intéressées et ça je pense que c'est un bon thème de coopération et donc au fond, je reste un peu. je suis un, un, un furieux séguiniste donc je j'ai j'ai une forme de prudence quand même par rapport à un certain nombre de coopération européenne mais là je dois bien avouer que sur Takuba. Il y a quand même une envie de faire et je pense qu'il faut qu'on l'entretienne et qu'on la fasse vivre, on la retrouve dans Atalante. La 2ème des choses qui me frappe beaucoup dans les différentes interventions et je pense que c'est important pour le ministre, et moi-même de le tenir comme un point d'étape. Dans la réarticulation de la présence française en Afrique, c'est au fond dans le creux de vos interventions, y en a pas un orateur qui au fond souhaite la même chose pour les missions que l'on donnera nos bases. Alors je vais commencer par le président Laurent qui veut les fermer. D'ailleurs, monsieur le président vous avez dit tout à la fois qu'il fallait être à l'écoute et dans le respect de la souveraineté de ces pays en même temps qu'il fallait fermer nos bases. Ça veut dire que lorsque les pays en question demande à ce que les bases prépositionnées reste ouverte et qu'elles accomplissent des missions, il faudrait quand même les fermer. Non mais je vous avez vous-même dit que vous êtes allés à la serpe. Donc je me permets de, de relever la la et en disant, vous voyez bien que les choses sont plus complexes et que dire on les ferme c'est c'est pratique mais enfin au fond c'est un peu rapide et que ça ne couvre pas l'ensemble des besoins. Inversement, pour d'autres, monsieur le sénateur, qui dit que moi je sais que vous relayer des préoccupations que vous entendez sur le terrain, mais les forces armées ne saurait avoir des missions. Comparables à celles des forces de sécurité intérieure des pays. Concernés en tout cas des pays qui nous accueille. Quand on a des intérêts économiques français dans un certain nombre de pays nos bases militaires sont là pour correspondre à des missions régaliennes prévus par des accords de défense, elles ne peuvent pas se mettre à intervenir pour protéger des intérêts économiques comme ça au quotidien sur une attaque qui relèverait d'une sécurité privée ou d'une sécurité de forces de sécurité intérieure. Donc ça je pense que c'est intéressant parce que de la fermeture des bases pur et simple du président Laurent ah et ce n'est pas du tout caricaturale. Je pense que ça ça revient le spectre de débats et de réflexion qui doit être le nôtre une intervention disant mais au fond monsieur miss, vous n'avez pas peur qu'avec la diminution de l'empreinte française nos intérêts économiques vont être davantage attaqué dans les pays concernés. Ah vous avez les deux, les deux grands opposés au fond des de positions qu'on a entendu dans l'hémicycle ce soir. Je pense que ça mérite d'y revenir en commission ou dans un autre moment parce que je pense qu'il faut pas qu'on se méprenne justement. Sur le rôle de nos bases et je me suis tenté de l'expliquer lors de du propos à la tribune. Faire croire qu'on peut faire sagittaire, avec la base de Djibouti, bah c'est vrai on l'a démontré récemment faire croire qu'on peut faire sagittaire, avec la base. Française au Sénégal. C'est faux, c'est faux aujourd'hui c'était faux, il y a 5 ans et c'était faux, il y a 10 ans. Les éléments français au Sénégal. Ce sont des éléments qui ne font que de la formation. Donc laisser à penser que la base militaire française au Sénégal peut faire la même chose qu'à Djibouti, où la même chose qu'à Abidjan c'est mentir à notre opinion publique ou c'est mentir à nos compétiteurs. oui quand le président de la République me donne mandat pour réarticuler la présence française en Afrique, je me suis aperçu quand même que j'ai beaucoup de même de bons connaisseurs des sujets militaires. Bah au fond on faisait passer une base pour l'autre. Non ce que sait faire la base projeté de Niamey où à la base projeté que nous avons. Par exemple au Niger ne correspond pas aux mêmes besoins militaires et au même contrat opérationnel que ce que nous savons faire au Gabon, le Sénégal et c'est pour ça que j'ai commencé par le Gabon, le Sénégal, parce que c'est l'héritage, qui montre bien qu'on n'a pas de fonction de combat. On a que des fonctions de formation et pour dire les choses, on a des fonctions de formation sur des besoins qui commence à devenir un tout petit peu passéistes ou en tout cas nous non satisfaisant par rapport aux besoins des forces armées des 2 pays en question je cas qui nous a qui nous accueille donc ça pour le coup je crois que c'est important et je je le ferais si présente comme on m'y autorise, peut être une nouvelle fois devant la commission en redisant bien les choses parce que sinon on entretient un flou évidemment on participe aussi aux narratif anti- français. Parce que faire croire que une base au Sénégal peut permettre de garder des intérêts politiques intérieures au Sénégal. C'est pas vrai parce que c'est ce qu'on dit parfois dans la presse. Donc je pense que là évidemment il faut. Y revenir de manière très précise dans la même veine, c'est mon 3ème point. Vous êtes nombreux à être avoir prononcé le fait qu'il fallait désormais être respectueux d'une véritable souveraineté. Des pays des États africains. Avec lequel nous entretenons des relations militaires, sécuritaires, le cas échéant, le ministre est revenu économique diplomatiques et moi évidemment j'adhère enfin je pense que peu de personnes assument dans cet hémicycle le fait que non il faut. Malmené bafouer la souveraineté des autres pays c'est pas le cas. Bon et puis pour autant très vite quand tu vos yeux se porte sur ce qui s'est passé au Mali. Vous en avez une lecture quand même qui est parfois très unilatérale. 13 expéditionnaire pour le coup et qui dit oui oui on s'est fait mettre dehors du Mali et cetera enfin je je l'ai dit un peu à la tribune. Enfin, que fallait-il faire et ce qu'il dit vous êtes restés trop longtemps, il fallait partir avant de se faire mettre dehors. Pourquoi pas, on ne sait toujours après mais enfin après tout je me dis. Certaines autres pays avec d'autres armées n'ont pris aucun risque, donc c'est sûr qu'on leur fait aucun reproche. Moi je ne nous appelle quand même une forme de solidarité aussi pour porter politiquement ce que font nos armées, on ne peut pas dire d'un côté ils ont été remarquables. On pense aux soldats et en même temps quand on fait les rétrospectives de ces missions ne pas assumer le portage politique j'ai cité le président Hollande tout à l'heure, je le redis ici, il fallait du courage au président de la République à l'époque pour engager les forces armées, à la demande du partenaire malien et d'expliquer devant l'opinion publique et la nation française de ce pourquoi il fallait le faire, bon il faut le redire. Et je pense que c'est notre honneur justement que de de laisser tomber toute forme de clivages politiques et de redire et de porter politiquement le bilan des décisions qui ont été prises à l'époque. j'ai pris des notes sur ce qui s'est dit le le vide laissé par nos militaires a appelé d'autres compétiteurs. Ça a été dit par certains. Par là-bas. Ça veut donc dire qu'il fallait rester alors contre l'avis même. Des de la de la junte. Malienne. Donc ça veut dire qu'il fallait rentrer en conflit ouvert avec la junte malienne et et les forces maliennes bon je trouve que tout ça. Franchement et et beaucoup plus compliqué quand on commence à le à le creuser et donc au fond. Ben oui il faut assumer quelque chose, c'est que quand un pays nous demandent de l'aide, il faut accepter de dire oui ou non et moi je salue une fois de plus la décision du président Hollande d'avoir dit oui, même si je note au fond cancre d'autres aurait dit non hein c'est ce qu'il faut quand même comprendre parfois dans sa zone d'intervention. Et que une fois qu'on a dit oui et bah, on ne sait pas toujours où est-ce que ça nous mène parce que parfois il y a un certain nombre d'événements politiques internes soit démocratique soit non démocratique qui n'était pas prévu et qui pour autant ne viennent pas effacer le risque terroriste et c'est quand même là aussi l'autre point sur lequel on n'est pas suffisamment revenu ce soir tout le monde l'a mentionné mais une fois de plus je l'ai dit, il devient endogène. Il est de nature différente. Il perles de plus en plus Moins homothétiquement quelque sorte qu'en 2013 2014 2015 et années suivantes et que donc, par définition il nécessite aussi un traitement militaire qui est d'une autre nature donc je pense que sur la question. de la vraie souveraineté. Du rôle de Barkhane. D'une, un accompagnement politique de la fin. Ben oui enfin pour ça il faut être deux. On peut pas dire qu'il faut faire à la place de ou faire à côté de et ne pas en tirer les conclusions en tout cas je le dis parce que je trouve que le procès devient facile si c'est pas le procès des forces armées, vous ne l'avez pas fait ce soir dans cet hémicycle enfin d'autres dans un autre hémicycle de l'autre côté de la Seine, ça s'est vu ces 15 derniers jours donc je le dis encore ici et puis même sur le volet politique. C'est pas une affaire de TP et d'argent que pour le Quai d'Orsay que de dire qu'à un moment donné, si la junte malienne préfère Wagner aux forces armées de la République française, c'est peut-être pas de la faute de Paris mais tout simplement la faute de la junte malienne. Je pense qu'on peut le dire aussi simplement que ça et ce n'est pas forcément donner un bon point, au président de la République ou à son gouvernement en le disant c'est juste tout simplement défendant les intérêts de la France. Ça me semble. Plein de bon sens que je dis mais je voulais quand même le redire parce que ça va mieux en le disant, voilà, je ne suis pas plus long. Ce que je retiens c'est que je pense qu'il faut une approche plus transparentes des missions que nos bases peuvent avoir à l'avenir. Je vais continuer, moi. À discuter avec les, les différents représentants et les différents homologues des pays concernés. On a un mouvement qui avance bien sûr un certain nombre de de base notamment sur des catalogues de formation qui serait nouveau, je pense que dès les prochaines cohortes de nos écoles sur le territoire national l'année prochaine on sera capable de vraiment de manière significative ré-accueillir beaucoup. D'élèves officiers ou élève sous-officiers venant de de ces écoles. Je pense que nous sommes en train de prendre du retard sur le spatial sur le cyber ou sur les drônes dans l'accompagnement de ces armées et qu'il nous faut désormais mettent les bouchées doubles. Autant de sujets très concrets qui nous fait un agenda d'influence par le concret et qui permet à la fois de lutter contre le terrorisme en même en même temps aussi de honorer notre parole parole que nous avons donné maintenant il y a plusieurs décennies parfois par des accords de défense. Je reste persuadé que le nord de la France, c'est de respecter la parole donnée lors de ces accords. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Ministre. Mes chers collègues, je vais lever la séance, notre prochaine séance aura lieu le mercredi 7 juin. À 15h pour les questions d'actualité au gouvernement. La séance est levée.